Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 4 novembre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. Mes chers collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation de la commission de l'administration du Sénat de la République tchèque, conduite par la vice-présidente du Sénat, Mme Jitka Seitlová.

demain. Cette visite intervient à la veille de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, laquelle comprendra un important volet parlementaire, notamment au Sénat. Elle sera suivie par la présidence de la République tchèque au second semestre. C'est dire toute l'importance des échanges entre nos deux assemblées. En vous souhaitant un séjour fructueux, mesdames, messieurs, je formule le voeu que votre visite contribue au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui lient la France et la République tchèque, ainsi que le Sénat français et le Sénat de la République tchèque. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2022

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chère Catherine Deroche, madame la rapporteure générale, chère Élisabeth Doineau,

la sécurité sociale de ce quinquennat. Mais s'il est le dernier, il n'en est pas le moindre, et nous n'allons pas relâcher nos efforts maintenant, bien au contraire, car il y a encore de beaux projets et de belles conquêtes Vous connaissez la situation des comptes sociaux. C'est peu dire qu'elle a déjà été meilleure, et c'est avec une petite pointe de nostalgie que je rappelle qu'il y a à peine deux ans, nous étions très proches d'un équilibre si longtemps espéré et attendu. Une pandémie mondiale est passée par là. Elle a exigé de notre part une action publique très ambitieuse et une intervention de l'État à des niveaux jamais atteints. Parce que, oui, l'État social a répondu présent pour offrir la meilleure protection possible à tous les Français, aux soignants comme aux soignés, aux travailleurs comme aux retraités, aux entreprises comme aux salariés, aux parents comme aux enfants, aux biens portants comme aux malades. Au début de ce quinquennat, nous voulions poser les fondations de l'État-providence du XXI siècle. Ce projet politique s'est heurté à la force des circonstances et d'un choc historique sans précédent. Aujourd'hui plus que jamais, nos systèmes de solidarité et de santé sont regardés pour ce qu'ils sont les piliers d'une grande Nation dans laquelle les hôpitaux accueillent chacun, quel que soit son prénom, quel que soit son statut et quels que soient ses revenus. Notre protection sociale n'est pas qu'une grande machine assurantielle ou un agrégat de tableaux sophistiqués et de mesures techniques accessibles à un cercle restreint de spécialistes. Elle est encore moins un musée que l'on regarderait avec une certaine nostalgie. Notre protection sociale est une réponse aux défis d'aujourd'hui et de demain, qui relèvent non pas de ceux qui agitent les plateaux de télévision et ne concernent que peu la vie réelle des Français, mais de ceux qui se manifestent parfois dans l'urgence, souvent dans la détresse, et toujours dans les morsures du quotidien. Nous ne parlerons pas d'autre chose dans les jours et les semaines qui viennent, et c'est tant mieux. Mesdames, messieurs les sénateurs, si la crise sanitaire a engendré 33 milliards d'euros de dépenses exceptionnelles

C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai demandé au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) de réfléchir à l'articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaire. J'observe que cette question fait d'ores et déjà couler beaucoup

Par ailleurs, et cela n'aura échappé à personne, du moins je l'espère, nous avons engagé un réinvestissement massif dans notre système de santé grâce au Ségur de la santé : 12,5 milliards d'euros en 2020, dont 10 milliards d'euros pour revaloriser les carrières de celles et ceux qui soignent, et 2,5 milliards d'euros pour l'investissement matériel. Contrairement à ce que j'entends parfois, et je tiens là encore à être très clair, aucune économie ne sera faite sur le dos de l'hôpital public. Croyez bien que je n'élude pas les difficultés, et même le malaise qui traverse

envergure, qui vont durablement transformer l'offre de soins dans les territoires, permettre de moderniser les structures et redonner du sens au quotidien de celles et ceux qui soignent.

Nous voulons également tirer profit de ce qui a fonctionné pendant la crise et pérenniser des innovations qui semblaient hier audacieuses et qui sont désormais bien présentes dans la vie des Français et des professionnels de santé. Je pense par exemple au numérique en santé, avec la téléconsultation et le télésoin : je le rappelle, nous sommes passés en quelques jours de plusieurs milliers à 1 million de téléconsultations par semaine durant la crise.

comme celle d'apporter des réponses concrètes à nos concitoyens en perte d'autonomie. En effet, il faut regarder en face la réalité du grand âge et prendre à bras-le-corps ce bouleversement démographique sans précédent. française, les sociétés européennes dans leur ensemble vieillissent. Nous le savons, il ne s'agit pas là d'une projection vague et abstraite, c'est déjà le cas ici et maintenant. Dans toutes les familles de France et de Navarre, c'est un sujet de préoccupation, parce qu'un parent ou un grand-parent qui perd son autonomie, c'est toute une organisation à penser ou à repenser.

2022 prévoit donc une réforme de l'autonomie, notamment pour renforcer la lisibilité et la qualité de l'offre à domicile, parce que pouvoir vieillir chez soi, bien vieillir chez soi est l'une des premières aspirations de nos aînés.

pérenne. Le Gouvernement propose notamment d'instaurer et de financer un tarif national de 22 euros par heure d'intervention, c'est-à-dire un niveau de financement public minimum, pour tous les services d'aide à domicile, ce qui représente un investissement de 240 millions d'euros dès 2022. Avec le Ségur de la santé, d'une part, l'agrément de l'avenant n° 43 à la convention collective de la branche de l'aide à domicile, d'autre part, ce sont plus de 2,8 milliards d'euros qui seront alloués chaque année au financement de revalorisations salariales.

Les déserts médicaux, que l'on nomme de manière plus administrative et moins brutale les « zones sous-denses », constituent un problème ancien, voire très ancien. Aussi loin que je me souvienne, la démographie médicale était déjà au coeur des préoccupations lors de mes études de médecine. Là encore, les députés ont formulé des propositions qui doivent permettre un accès aux soins plus direct et plus simple, et avec un niveau élevé de qualité, dans tous les territoires. Je pense ici à la prise en charge des consultations auprès des psychologues en ville, à la suite des annonces du Président de la République dans le cadre des assises la prise en charge intégrale, pour les jeunes hommes de moins de 25 ans, d'une consultation longue en santé sexuelle, afin de mobiliser les garçons autour des thématiques de santé sexuelle, notamment sur le choix d'une contraception adaptée, l'encadrement renforcé des centres de santé, en particulier pour les soins dentaires et optiques, afin de garantir des prestations de qualité. Qui dit accès aux soins dit également accès aux traitements. Si cela passe par un meilleur financement de l'innovation et une meilleure sécurité d'approvisionnement en médicaments, il faut aussi responsabiliser les laboratoires, en continuant à baisser les prix sur les produits les plus amortis, afin d'éviter les phénomènes de rente, ou en étant plus exigeant sur les ruptures de stock.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nos débats seront l'occasion d'aller encore plus loin dans beaucoup de domaines et sur des sujets dont la crise a prouvé qu'ils étaient parfois d'une envergure insoupçonnée, comme c'est le cas, par exemple, de la santé mentale, dont nous n'avons jamais autant parlé. Je m'en félicite d'ailleurs, parce qu'elle a trop longtemps été le parent pauvre de nos politiques de santé.

aussi avoir une certaine idée de sa protection sociale, hier, aujourd'hui et demain. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, cher Olivier, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure générale, mesdames, messieurs les rapporteurs,

sociale. Ces chiffres contrastent fortement avec les ambitions que nous nourrissions avant la crise sanitaire, quand le retour à l'équilibre de la sécurité sociale était proche et que l'amortissement de la dette sociale avait vocation à s'arrêter en 2024. Ainsi, après révision, le déficit du régime général de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) devrait s'établir à 33,5 milliards d'euros en 2021, à 20,4 milliards d'euros en 2022, et dépasser encore 11 milliards d'euros en 2025. Par rapport aux agrégats figurant dans le texte initial, qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale, le déficit serait ainsi diminué de 1,1 milliard d'euros en 2021, de 1,2 milliard d'euros en 2022 et de 2,2 milliards d'euros en 2025.

Tous les Français sont conscients, je le crois, de l'immense effort que notre système de santé a fourni et continue de fournir pour lutter contre la crise sanitaire et les protéger. Cet effort est bien entendu d'abord celui des soignants, que je tiens encore à saluer. C'est également un effort financier d'une ampleur colossale. Je rappellerai quelques chiffres 135 millions, c'est le nombre de tests de dépistage que nous avons réalisés, soit davantage que tout autre pays en Europe ; 4,7 milliards d'euros, c'est l'estimation du coût de notre campagne vaccinale, que je considère toujours comme le meilleur investissement qui soit, non seulement pour la santé de nos concitoyens, mais également pour le redémarrage de notre économie. La crise sanitaire a rendu plus concrète que jamais la raison d'exister de la sécurité sociale : protéger les Français. Ne jamais prendre cette mission comme acquise, chercher continuellement à mieux protéger les Français, cela fait partie des objectifs que nous nous sommes fixés durant ce quinquennat. Je ne reviendrai pas en détail sur chacune des avancées de ce quinquennat en matière de droits sociaux. Je citerai seulement les principales d'entre elles : le déploiement du dispositif « 100 % santé », une réforme qui a changé le quotidien de millions de nos concitoyens

sécurité sociale présentés durant ce quinquennat ont également été l'occasion de traduire un autre fil rouge de notre action, sur lequel je souhaite revenir : je veux parler de la revalorisation du travail et de notre engagement en faveur de l'emploi et de la croissance. d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en un allégement pérenne de charges sociales de plus de 23 milliards d'euros et supprimé les cotisations salariales chômage et maladie, soit un effort supplémentaire de 6 milliards d'euros en faveur des actifs. Nous avons supprimé les cotisations sociales sur les heures supplémentaires, par ailleurs défiscalisées. Nous avons enfin étendu les allégements généraux à l'ensemble des contributions sociales, afin qu'il n'y ait plus de cotisations ou de contributions patronales au niveau du SMIC. Cette politique en faveur de la croissance, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été une constante de notre action. Nous l'avons poursuivie sous une autre forme en octroyant des aides massives aux entreprises et aux salariés en activité partielle durant la crise sanitaire, et ce en un temps record. Nous l'avons prolongée en déployant France Relance, un plan de relance de l'activité inédit de 100 milliards d'euros, qui servira notamment

Cette politique porte ses fruits. Nous avons ainsi relevé nos prévisions de croissance de 6 à 6,25 % pour 2021, ce qui conduit à la révision de la trajectoire pluriannuelle que je viens de vous détailler. Comme pour le projet de loi de finances, je précise que, si la croissance constatée

ailleurs un levier majeur de simplification pour les entreprises qui n'auront plus, à terme, qu'un seul interlocuteur au titre des cotisations sociales. Vous aviez adopté une trajectoire ambitieuse d'unification du recouvrement social dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Certains de ces jalons ont pu ou pourront être aménagés, afin de tenir compte des effets de la crise sanitaire et de sécuriser les transferts. Ainsi, le transfert des cotisations collectées par l'Agirc-Arrco sera amorcé en 2022 par un pilote ; sa mise en oeuvre pleine et entière n'interviendra, quant à elle,

Je souhaiterais évoquer rapidement deux autres mesures de transformation prévues dans ce texte. Nous vous proposons de généraliser le versement en temps réel des aides fiscales et sociales du secteur de l'aide à domicile, à commencer par le crédit d'impôt au titre des services à la personne.

À partir de 2023, une fois les conventions de partenariat conclues avec les conseils départementaux, ce sont les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, ou de la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui entreront dans le dispositif ; enfin, en 2024, cette généralisation sera élargie à la garde d'enfants. Cette réforme simplifiera la vie de millions de nos concitoyens qui doivent aujourd'hui avancer le montant de leur crédit d'impôt. Elle contribuera à accompagner le virage domiciliaire et l'essor du secteur des services à la personne et de l'aide à domicile. Elle simplifiera le développement du travail déclaré et favorisera ainsi l'ouverture des droits sociaux associés aux salariés concernés.

de neutraliser les effets de la crise, de faciliter l'ajustement des échéances de cotisations sociales par les travailleurs indépendants eux-mêmes en fonction des revenus perçus et de moderniser le statut de conjoint collaborateur.

Nous avons également besoin d'un pilotage unifié des finances sociales, ce qui implique, au vu du déficit global, de ne pas considérer les éventuels excédents isolés comme des marges de manoeuvre, mais de renforcer la solidarité interbranches. Nous devrons évidemment poursuivre les réformes structurelles lorsque les conditions seront réunies. après des exercices forcément exceptionnels, nous devrons renouer avec un pilotage rénové des dépenses d'assurance maladie, qui ne soit pas incompatible avec nos objectifs en matière de santé publique, mais qui garantisse au contraire une utilisation plus juste des contributions des Français à notre système de protection sociale. 2022 ne solde donc pas l'ensemble des sujets. Il clôt toutefois un quinquennat de transformation de notre système social et d'avancées en faveur d'une meilleure protection des Français. Dans ces temps difficiles, la sécurité sociale a de nouveau prouvé sa modernité. Il nous reste à faire en sorte collectivement de lui permettre de continuer, demain, à remplir sa mission de protection des Français.

le plus lourd déficit de l'histoire des comptes sociaux. J'y reviendrai simplement à votre suite, messieurs les ministres, pour souligner une nouvelle fois que, dans une période de crise d'une très grande violence, la sécurité sociale a su pleinement jouer son rôle en aidant les Françaises et les Français, sanitaire de la crise que de son volet social. Le Sénat et sa commission des affaires sociales ont d'ailleurs pleinement soutenu cette démarche, même si nous avons pu regretter, à raison, de ne pas avoir été consultés un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

je retiendrai surtout la prolongation de neuf ans de l'existence de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), notamment pour éponger quelque 92 milliards d'euros au titre des déficits anticipés à partir de 2020. Pour l'année 2021, l'amélioration des comptes n'est que peu sensible, malgré une vigoureuse reprise économique et la forte diminution du recours à l'activité partielle.

Certes, la prévision de solde est pratiquement identique à ce que prévoyait la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Mais c'est de l'ordre de l'apparence, puisque cela découle d'une augmentation des recettes comme des dépenses d'un peu moins de 12 milliards d'euros

Là encore, messieurs les ministres, la consultation du Parlement en cours d'exercice aurait été préférable. À l'issue de ces deux années bouleversées par la crise, c'est bien l'évolution des finances sociales qui se joue dès le PLFSS pour 2022. Or, mes chers collègues, de ce point de vue, je ne peux vous cacher les inquiétudes que m'inspire ce texte. Certes, pour l'exercice à venir, le déficit de la sécurité sociale devrait s'améliorer assez nettement, pour revenir à 22,6 milliards d'euros au niveau des Robss et du FSV, ce qui reste considérable. Cette amélioration, qui pourrait d'ailleurs être encore plus forte du fait de la révision des hypothèses macroéconomiques, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre Dussopt, n'est due qu'à l'embellie économique. Ce sont bien les recettes, tirées par la hausse du PIB et de la masse salariale, qui comblent en partie le trou des années 2020 et 2021. En revanche, aucune mesure nouvelle, notamment en dépenses, ne contribue à cette amélioration. L'annexe 4 du PLFSS montre d'ailleurs bien que les mesures nouvelles dégradent légèrement le solde. Je peux comprendre ce choix pour l'année à venir, non seulement en raison des échéances électorales, mais aussi parce qu'en sortie de crise la France reste fragile d'un point de vue économique et social. Dans ce contexte, il importe sans doute de ne pas briser l'élan, d'autant que nul ne sait ce que nous réserve l'épidémie de covid-19 à l'avenir. C'est sur l'avenir un peu plus éloigné que se porte l'essentiel de mes inquiétudes. En effet, comme vous le savez, le PLFSS présente l'originalité de comprendre une annexe à la fois « littéraire » et financière relative aux quatre prochaines années, ce qui peut évidemment inclure l'effet de mesures nouvelles à venir. Or, messieurs les ministres, cette annexe ne dessine aucune stratégie de retour à l'équilibre pour les quatre années à venir, après la crise actuelle. Bref, il n'y a aucun signe de « dégrisement » après le « quoi qu'il en coûte En conséquence, malgré le rebond économique de 2021 et 2022, la trajectoire des comptes de la sécurité sociale tranche nettement avec ce qui a été observé lors de la crise financière de 2008. le décrochage initial est plus élevé, mais surtout le déficit des Robss et du FSV devrait atteindre un plateau dès 2023, à un niveau d'une quinzaine de milliards d'euros littéralement insoutenable pour la sécurité sociale. Cette trajectoire contraste nettement avec le chemin suivi après la crise financière de 2008, dans un contexte de langueur économique sur une plus longue période. Pour ces raisons, la dette sociale n'apparaît pas maîtrisable.

Surtout, la poursuite de l'accumulation de déficits importants après 2022, actée par le Gouvernement, conduirait à dépasser ce plafond de plus de 51 milliards d'euros d'ici à 2025. Bien entendu, en l'absence de stratégie de retour à l'équilibre, il n'y a aucune raison de croire que les déficits se résorberont comme par magie à partir de 2026.

Au total, la trajectoire financière proposée par le Gouvernement semble réellement hypothéquer notre capacité collective à léguer notre système de protection sociale aux générations futures. Face à cette situation, notre commission a pris ses responsabilités et choisi d'afficher un message clair. D'une part, en rejetant le rapport annexé, dont le fond restera inchangé même avec les éventuels amendements que le Gouvernement pourrait présenter. D'autre part, en formulant plusieurs propositions concrètes destinées à envoyer un message de responsabilité financière sans casser la reprise en cours. Ces propositions se déclineront autour de trois axes. consiste à ne faire assumer à la sécurité sociale que les coûts lui incombant. Je pense notamment à l'explosion du budget de Santé publique France et à la dette hospitalière, à assurer, avec notre rapporteure de la branche maladie, Corinne Imbert, et dans la continuité de nos propositions en loi organique, un meilleur contrôle du Parlement sur les multiples dotations que la sécurité sociale, en particulier cette branche maladie, verse à différents organismes. Le troisième consiste à avancer, avec notre rapporteur de la branche vieillesse, René-Paul Savary, une proposition qui associera les partenaires sociaux tout en affichant la nécessité d'évolutions paramétriques en matière de retraite. En somme, messieurs les ministres, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a fait le choix de la cohérence, afin de préserver à long terme la solidité de notre modèle social. Soyons conscients que seule une sécurité sociale avec des comptes en ordre nous permettra d'offrir la même protection à nos enfants et de faire face à la prochaine crise.

les ministres, nous paraît particulièrement préoccupante. Force est de constater que les revalorisations du Ségur de la santé ne sont pas financées et qu'en présentant une perspective de déficit à hauteur de 15 milliards d'euros pour 2025, le Gouvernement met l'assurance maladie dans une situation de grande fragilité. Quel avenir assurons-nous au financement de notre système de santé avec pas moins de 63 milliards d'euros de déficits cumulés entre 2021 et 2025 ? La Cades paiera sans doute L'Ondam devrait atteindre l'an prochain 236,3 milliards d'euros, soit, en définitive, un montant en très léger repli par rapport à la rectification pour 2021. Mais, hors dépenses liées à l'épidémie de covid-19, il sera en progression de 3,8 %. C'est une dynamique particulièrement forte. Vous nous répondrez que l'Ondam pour 2022 est ambitieux et revendiquerez un effort sur le médicament et une absence d'économies sur l'Ondam hospitalier. Soit ! Pourtant, ce niveau de dépenses record dont vous vous réjouissez nous semble en décalage criant avec la réalité que nous constatons tous dans nos territoires des situations parfois alarmantes, avec des services d'urgence hors d'état de marche, ainsi qu'un profond et préoccupant malaise de certaines professions de santé- comment ne pas citer les sages-femmes, ou encore les internes articles sont rattachés à la branche maladie. N'ayant pas le temps de les détailler, je me limiterai à quelques observations. S'agissant de l'hôpital, les dispositions proposées se bornent à des ajustements des réformes structurelles du financement de la psychiatrie, des soins de suite et de réadaptation et des urgences, rendus nécessaires par la crise sanitaire. Sur le volet des produits de santé, le PLFSS pour 2022 se revendique comme celui de la mise en oeuvre des mesures arrêtées par le Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) de 2021 et celles du plan Innovation Santé 2030, qui en découle. Si l'article 36, avec le nouveau dispositif dit d'« accès direct » au médicament, et l'article 38, traitant de la prise en compte de l'empreinte industrielle dans la fixation du prix, nous paraissent bienvenus, nous sommes plus réservés sur leur mise en oeuvre concrète. Dans le champ du dispositif médical, je me félicite de la création, à l'article 24, d'un régime de prise en charge de droit commun des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance et, à l'article 33, d'un accès à une prise en charge anticipée pour ceux de ces dispositifs qui présenteraient un caractère innovant. Concernant les soins de ville, le PLFSS comporte plusieurs articles qui visent à faciliter l'accès à certains soins dispensés par des auxiliaires médicaux, en supprimant la prescription médicale préalable. Sur ce point, disons-le, il ne remplit pas son rôle. Les dispositions que vous y avez inscrites, messieurs les ministres, comme les articles additionnels adoptés à l'Assemblée nationale ont transformé ce texte en une loi de santé au rabais, ficelée à la hâte avant la fin de votre mandat, Ce n'est pas satisfaisant sur la forme : c'est un dévoiement du PLFSS. Ce n'est pas non plus satisfaisant sur le fond : ces mesures, qui répondent parfois à de réelles lacunes dans nos territoires, méritaient une vraie concertation avec l'ensemble des professionnels concernés, d'autant que certains des dispositifs envisagés risquent de mettre à mal, sur le long terme, le rôle du médecin traitant et le principe même de parcours de soins coordonnés. Très juste ! Enfin, dans le domaine de la prévention, le PLFSS comprend une série de mesures disparates, consistant essentiellement à généraliser ou prolonger des expérimentations, dont la commission partage l'intention globale, même si elle en regrette parfois le manque d'ambition. Telles sont en quelques mots, mes chers collègues, mes principales observations sur la branche maladie et les dispositions la concernant, que la discussion des articles doit désormais

à l'heure où nous abordons l'examen du dernier PLFSS du quinquennat, je ne peux m'empêcher de repenser à la grande réforme du système de retraite promise par le candidat Emmanuel Macron en 2017. Nous allions voir ce que nous allions voir ... Nous n'avons toujours rien vu ! Pendant ce temps, les perspectives de retour à l'équilibre de la branche vieillesse ne cessent de s'éloigner et relèvent davantage de la chimère que du champ des possibles. Après la forte dégradation, en 2020, de la situation financière de la branche, dont le déficit a atteint 7,4 milliards d'euros sous l'effet de la crise sanitaire, l'amélioration de la conjoncture économique ne devrait pas permettre de ramener le solde à son niveau de 2019, tant s'en faut. Ainsi, grâce à la progression du produit des cotisations sociales, liée à la fois à l'accroissement de la masse salariale et à la régularisation des cotisations reportées des travailleurs indépendants, le déficit de la branche vieillesse reculerait à 6,4 milliards d'euros en 2021 et à 5,2 milliards en 2022. Ajoutons que cette tendance ne durerait pas au-delà de 2022. Dès 2023, en raison de la vigueur de l'inflation et de la poursuite du vieillissement démographique, le déficit de la branche se dégraderait de nouveau, pour atteindre 10 milliards d'euros d'ici à 2025. À mesure que se profile ce sinistre horizon, qui remet gravement en cause la confiance des jeunes générations en la capacité du système de retraite à leur garantir une pension en contrepartie des cotisations versées tout au long de leur carrière, pour la cinquième année consécutive

relatives à l'assurance vieillesse, comme la validation de trimestres de retraite par les travailleurs indépendants frappés par la crise, la possibilité de racheter des trimestres pour certains travailleurs indépendants, dont les cotisations n'ont pas été appelées pendant de nombreuses années, ou encore l'extension de la retraite progressive aux cadres en convention de forfait en jours, ce PLFSS ne contient aucune mesure de redressement des comptes de la branche vieillesse. Comme chaque année, la commission prendra donc ses responsabilités- remercie, madame la rapporteure générale, de l'avoir souligné -en proposant à la représentation nationale d'adopter, en vue d'un retour à l'équilibre à l'horizon de 2030, les seules mesures envisageables compte tenu de notre refus catégorique du recours à la diminution des pensions ou à l'augmentation des cotisations. Réaffirmant notre attachement au paritarisme, nous proposons de confier aux partenaires sociaux, réunis dans le cadre d'une conférence de financement- nous n'avons rien inventé -, la charge de formuler des propositions en ce sens en recourant à divers leviers. Dans le cas où cette conférence ne parviendrait pas à trouver un consensus, nous ne souhaitons pas, les ajustements paramétriques qui nous paraissent nécessaires entreraient en vigueur dès 2023. Il s'agit, d'une part, du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans dès la génération 1966 et, d'autre part, de l'accélération de la mise en oeuvre de la réforme Touraine, de façon à ce que la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein soit portée à 43 annuités à compter de la génération 1966, au lieu de la génération 1973. En somme, mes chers collègues, la question fondamentale qui se présente à nous est la suivante voulons-nous faire peser sur nos enfants et nos petits-enfants le poids de la dette qui s'accumule jour après jour, à défaut de trouver le courage de mener enfin une réforme difficile, mais indispensable ? Laisser filer plus longtemps les déficits reviendrait à porter atteinte au principe même de répartition, fondé sur la solidarité entre les générations. Or qui dit solidarité, dit aussi équité : une génération ne doit jamais se trouver contrainte à payer les frais de l'incapacité des générations précédentes à assumer leurs propres responsabilités.

la branche famille retrouverait l'équilibre en 2021 avec un solde de 1,2 milliard d'euros. Le rétablissement des recettes de la branche serait porté par la reprise économique, tandis que les dépenses augmenteraient légèrement. Pour 2022, la situation de la branche continuerait à s'améliorer avec un excédent de 1,7 milliard d'euros. Si l'on peut se réjouir de ces perspectives financières rassurantes, le doute est permis quant au bon emploi des excédents retrouvés. Je ne peux ainsi cacher ma déception de voir la branche famille faire l'objet, une fois encore, de si peu de mesures dans le PLFSS, alors que la politique familiale dans notre pays a besoin d'un renouveau. Toutefois, les quelques dispositions proposées vont dans le bon sens, et c'est pourquoi la commission vous proposera de les adopter. La systématisation de l'intermédiation financière des pensions alimentaires constitue sans aucun doute l'avancée la plus importante. Elle parachève le mouvement de réforme visant à lutter contre les impayés des pensions alimentaires, en s'attaquant au problème à la racine. En 2019, nous avions voté en faveur du recours à l'intermédiation lorsqu'elle est mentionnée dans le titre exécutoire fixant la pension alimentaire ou lorsqu'un des parents demande sa mise en place auprès de sa caisse d'allocations familiales. L'article 49 propose d'aller plus loin en rendant applicable l'intermédiation de la créance alimentaire dès l'émission du titre exécutoire. Par dérogation, les parents pourront refuser conjointement ce dispositif, sauf si le parent créancier ou l'enfant a été victime de menaces ou de violences volontaires commises par le parent débiteur. La commission vous propose, mes chers collègues, d'adopter cet article, qui permettra de réduire l'insécurité financière des familles victimes d'impayés, notamment les familles monoparentales. La commission a également accueilli favorablement l'article 49 , qui simplifie les modalités de calcul et de revalorisation de la prestation d'accueil et de restauration scolaire versée dans les départements et collectivités d'outre-mer. Alors que les montants de la prestation ont été injustement gelés depuis plusieurs années, il est notamment proposé que sa revalorisation annuelle soit désormais indexée sur l'inflation. D'autres dispositions renforcent l'accès aux droits par l'échange de données entre organismes et administrations ou bien par une lutte accrue par les organismes débiteurs de prestations familiales contre le non-recours. Ces dispositions, qui correspondent largement aux pratiques déjà en vigueur, ne posent pas de difficultés de fond, sous réserve de quelques ajustements que je proposerai. Enfin, l'article 49 vise à décaler l'entrée en vigueur du tiers payant pour le complément de libre choix du mode de garde (CMG) accordé aux parents ayant recours à une structure pour la garde de leurs enfants. C'est avec regret- je l'ai déjà souligné en commission -que je constate l'impossibilité technique de déployer le tiers payant dès janvier prochain et la nécessité d'adopter cet article. Ainsi, je ne formule pas d'opposition sur les mesures proposées dans ce texte. Je constate en revanche que le Gouvernement n'enclenche pas la relance de la politique familiale dont notre pays a tant besoin au vu de sa natalité déclinante. De 2012 à 2019, le nombre annuel de naissances dans l'Hexagone est passé de 790 000 à 714 000. La remise en cause de notre modèle de politique familiale a sa part dans cette chute de la natalité. Introduite en 2015, la modulation du montant des allocations familiales selon les ressources du foyer a brouillé la lisibilité de notre système, en assignant un objectif redistributif à une prestation universelle. Il me semble nécessaire et urgent de revenir sur cette modulation. C'est pourquoi je déposerai prochainement une proposition de loi en ce sens. Le renouvellement des générations est le meilleur investissement pour l'avenir. Tout notre système de sécurité sociale, dont nous débattrons cette semaine, repose sur une démographie dynamique. Il convient donc de ne pas le mettre en difficulté

après la brutale dégradation du solde de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire, celui-ci revient en territoire positif pour l'année 2021. La branche serait ainsi excédentaire de 676 millions d'euros, tous régimes confondus, la reprise économique ayant tiré vers le haut la masse salariale sur laquelle sont assises les cotisations versées par les employeurs, ce que n'a pas annulé l'augmentation mécanique des accidents du travail au sortir de l'année 2020. Une augmentation de cet excédent est prévue pour l'an prochain, conduisant les capitaux propres de la branche à culminer à plus de 5 milliards d'euros à la fin de 2022. À long terme, toutes choses égales par ailleurs, les recettes de la branche AT-MP restent donc structurellement plus dynamiques que ses dépenses. Cela signifie que les prestations fournies par la branche ne sont pas au niveau de la contribution demandée aux employeurs. L'extension du périmètre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) aux médicaments antiparasitaires vétérinaires et l'égalisation des conditions de reconnaissance des maladies professionnelles dans le secteur agricole entre l'outre-mer et l'Hexagone n'auraient qu'un impact financier extrêmement limité pour 2022 et les années à venir, de l'ordre du million d'euros. Si je souscris à ces mesures, je déplore le déploiement tardif du FIVP : celui-ci n'est intervenu qu'à la fin de l'année 2020.

Il est d'autant plus notable- ou dommageable -que la principale mesure financière de ce projet de loi concerne l'augmentation de 100 millions d'euros du transfert effectué par la branche AT-MP au bénéfice de la branche maladie du régime général, au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce versement atteindrait 1,1 milliard d'euros, ce qui représente près de 8 % de l'objectif de dépenses pour la branche ! Cette augmentation fait suite au dernier rapport de la commission qui évalue, tous les trois ans, le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des AT-MP, en se fondant sur des études épidémiologiques et, surtout, statistiques. Ce coût, selon le rapport de juin 2021, serait compris entre 1,2 et 2,1 milliards d'euros. Le Gouvernement s'est fixé pour horizon d'atteindre la fourchette basse de l'estimation, soit 1,2 milliard d'euros, dès 2023. Le maintien de ce transfert à un niveau aussi élevé, s'il se fonde sur les travaux de la commission d'évaluation, est avant tout le fruit d'un choix politique. Il laisse entendre qu'aucun progrès n'a été accompli sur la question de la sous-déclaration, ce qui est faux. Plusieurs des recommandations du rapport de 2017 ont été mises en oeuvre et celles du rapport de 2021 sont en passe de l'être. Tout porte plutôt à croire que ce versement, dont le montant est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation AT-MP et pèse donc sur les entreprises, sert principalement à contribuer au rééquilibrage de la branche maladie. Or, la cotisation AT-MP est censée responsabiliser les employeurs sur leur sinistralité, et non pallier les difficultés d'autres branches. J'observe que, si pendant les sept dernières années, lors desquelles le transfert à la branche maladie a été fixé à 1 milliard d'euros, ce versement avait pris pour référence la fourchette basse des estimations de la commission d'évaluation, soit près de 800 millions d'euros, il s'en serait suivi un gain moyen pour la branche d'un peu plus de 200 millions d'euros. Il conviendrait de les soustraire au 1,2 milliard que se propose d'atteindre le Gouvernement. La commission des affaires sociales a donc adopté un amendement tendant à maintenir le montant du versement pour 2022 à la branche maladie à 1 milliard d'euros. La différence pourrait judicieusement être utilisée pour financer des actions de prévention dans le cadre de la prochaine convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. En particulier, si un report de l'âge de départ à la retraite était mis en oeuvre, les conditions de travail des futurs retraités devraient leur permettre de partir à l'âge prévu en bonne santé, quand aujourd'hui de nombreux salariés en fin de carrière sont fréquemment en arrêt de travail. Si je ne méconnais pas les efforts que déploie la branche AT-MP en la matière, j'ai été alertée sur le fait que le capital de subventions attribuables aux été entièrement consommé dès avril de cette année, ce qui indique un problème d'offre par rapport à la demande de prévention. La branche pourrait donc, compte tenu de ces marges de manoeuvre financières, prévoir une augmentation enfin conséquente des dépenses de prévention, dans la lignée de la loi votée cet été, et poursuivre dès que possible l'ajustement à la baisse des cotisations, en cohérence avec la baisse tendancielle, bien qu'inégale selon les secteurs, de la sinistralité. mes chers collègues, je vous invite à vous prononcer en faveur de l'objectif de dépenses de la branche, fixé à 14,1 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base pour 2022. La parole

cette nouvelle étape de l'histoire de la sécurité sociale est à l'heure d'un premier bilan. Il est bien mince. Aucune conséquence n'a été tirée de la création d'une nouvelle branche qui comprend, comme l'an dernier, les dépenses de la Caisse nationale de solidarité

L'objectif de dépenses de la branche pour 2022 s'élève à 34,2 milliards d'euros, soit 800 millions d'euros de plus que le tendanciel de dépense. Cette somme, non négligeable, finance notamment deux nouveautés, que je salue. est l'extension des revalorisations salariales issues du Ségur de la santé aux agents de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents exerçant comme soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements financés au moins en partie par l'Ondam. un large pan du champ médico-social, mais pas son intégralité. Ces revalorisations successives, par cercles excentriques, de l'hôpital vers le secteur social sont incompréhensibles pour les personnels sur le terrain, voire pour l'administration elle-même. Encore un problème de méthode. Elles déstabilisent un secteur aux statuts très hétérogènes du fait de l'aspiration des professionnels par les services concernés par les revalorisations. Nombreuses sont les structures associatives qui sont aujourd'hui menacées de fermeture. Dans le secteur du handicap, l'alerte est extrêmement sérieuse.

De nouveau, une question de méthode se pose. En effet, il est regrettable que l'ensemble des acteurs du domicile n'aient pas été intégrés à cette réforme et que nous n'ayons pas profité de cette opportunité pour évoquer le mode mandataire, l'emploi direct et les prestataires de santé à domicile. Une « dotation qualité » de 3 euros financera des services s'engageant par contrat avec les départements à respecter certaines contraintes. C'est une avancée notable vers la rationalisation de l'offre et l'amélioration du financement de ces structures. Ces mesures, qui vont dans la bonne direction, illustrent les limites d'une méthode consistant à retoucher ce qui peut l'être en loi de financement, faute d'avoir pu transformer en loi la concertation pourtant bien engagée sur le grand la vision d'ensemble est quasi absente, la concertation préalable avec les professionnels ou les départements faible, mais la complexité s'accroît à chaque dispositif nouveau. Songez que les concours de la CNSA aux départements transiteront désormais par une dizaine de canaux différents À ces dispositifs d'intérêt variable, les députés ont ajouté, sur l'initiative du Gouvernement ou du groupe majoritaire, huit autres articles d'un intérêt, si je puis dire, plus variable encore. Je ne prendrai pour exemple que l'expérimentation d'une carte professionnelle pour les salariés du domicile, qui serait anodine si le climat n'était pas aussi tendu pour le secteur. La commission vous proposera de la supprimer. En 2003, la canicule avait donné lieu à la création de la CNSA, de la journée de solidarité et d'un plan pour le grand âge. Derrière ces dispositifs, quelques idées simples : l'engagement d'une réflexion stratégique sur l'autonomie une caisse à la gouvernance innovante ; la création de ressources nouvelles ; un début de vision pluriannuelle. Dix-huit ans plus tard, après un traumatisme social au moins égal en intensité, que propose le Gouvernement ? La transformation, sans conséquences opérationnelles, de la CNSA en caisse de sécurité sociale, d'innombrables missions et groupes de travail dont peu d'enseignements sont tirés et quelques mesures nouvelles que je vous ai présentées. Ces efforts ne sont pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Pour maintenir les questions d'autonomie à l'agenda politique et qu'enfin des décisions de financement soient prises, la commission des affaires sociales vous propose d'institutionnaliser le dialogue entre les différents partenaires, sous la forme d'une conférence annuelle des générations et de l'autonomie, alimentant le travail du Parlement.

Au regard de ses effets sur nos finances publiques, la commission des finances a souhaité se saisir pour avis de ce texte. Cet avis porte principalement sur la trajectoire des comptes sociaux. Les finances de la sécurité sociale se trouvent aujourd'hui prises entre deux tendances contradictoires : la crise sanitaire a provoqué un effondrement sans précédent des comptes de la sécurité sociale, les mesures de confinement s'étant poursuivies dans la première moitié de l'année. Dans le même temps, la reprise économique, plus vigoureuse que prévu, vient améliorer les prévisions de recettes et de solde par rapport à celles qui étaient inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale de l'année dernière. Cette reprise économique, si elle est bien entendu une bonne nouvelle, ne doit pas faire oublier les risques majeurs qui pèsent aujourd'hui sur les comptes sociaux. Je préfère ainsi parler de « convalescence » des comptes sociaux s'il y a indéniablement une amélioration des indicateurs, les effets de la crise se font encore sentir, et elle continuera à marquer la trajectoire des finances sociales pour de nombreuses années à venir. En 2022, nous pouvons espérer que l'essentiel de la crise sera derrière nous. Cet optimisme se traduit dans les prévisions pour les comptes sociaux : le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) devrait être ramené à 21,6 milliards d'euros,

et c'est aussi le moment où nous devons nous interroger sur la trajectoire des comptes sociaux et leurs risques de dérives. En effet, il est possible désormais de mieux distinguer entre les augmentations de dépenses, qui visent à répondre immédiatement à la crise, et celles qui ont vocation à s'installer dans la durée. Les premières ne représentent pas une menace pour les comptes sociaux, contrairement aux secondes. À ce titre, laissez-moi citer un chiffre : il est estimé qu'à l'horizon 2024, le déficit du régime général et du FSV serait supérieur à 10 milliards d'euros. Ces déficits sont qualifiés par la Cour des comptes, dans son rapport du début d'octobre, de « permanents » ; c'est-à-dire qu'ils ne se résorberont pas, sauf mesures nouvelles ou « miracle » économique. L'amélioration des indicateurs économiques par rapport à ceux qui sont inscrits dans le PLFSS ne sera pas suffisante pour changer cet état de fait. Il demeurera toujours à partir de 2024 un déficit permanent et élevé. Or plus longtemps on maintiendra ce déficit, plus il sera difficile d'inverser la tendance et plus la perspective d'un retour à l'équilibre des comptes s'éloignera. Mais tout le problème est là : le projet de loi de financement de la sécurité sociale ne présente aucune mesure structurelle forte à même de rétablir la trajectoire des comptes de la sécurité sociale. Toutes les mesures de maîtrise des dépenses ne sont pas incompatibles avec la croissance économique ; certaines peuvent au contraire la favoriser. Je pense par exemple à la lutte contre la fraude sociale. La seule mesure présente dans le texte est une simplification marginale du processus de contrôle. La grande absente du projet de loi reste la réforme des retraites. En effet, quoique la branche vieillesse n'ait été que marginalement affectée par la crise, elle est aujourd'hui celle qui connaît l'évolution, en pourcentage, la plus inquiétante. plus inquiétante. Le déficit de la branche vieillesse devrait, en 2025, être plus de trois fois supérieur à celui de 2022. Nous sommes ainsi obligés de poser à nouveau la question de la gestion de la dette sociale. Le présent projet de loi de financement met en avant des déficits cumulés du régime général et du FSV supérieurs à 92 milliards d'euros pour la période 2020-2023. En outre, un déficit de 10 milliards d'euros est attendu pour l'exercice 2024. pour celui de 2025. Ces perspectives rendent irréaliste la prévision actuelle d'une extinction de la Cades aux environs de 2033. Il apparaît alors que le poids de la dette sociale est confié aux générations futures, ce que l'on cherchait pourtant à éviter avec la création de cette caisse en 1996. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission des finances a émis un avis défavorable sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Conformément aux promesses de 1945, il a protégé leurs revenus contre les aléas de l'existence- ceux-ci ont été nombreux au cours des deux dernières années -et a pris soin de leur santé dans un cadre solidaire. Nous attendons légitimement beaucoup de notre protection sociale, qui fait partie de notre bien commun. Mais le financement de ce bien commun n'a rien du miracle : il repose sur les ménages et les entreprises qui manifestent souvent, désormais, sous des formes diverses, une certaine lassitude à l'égard des prélèvements obligatoires. La crise sanitaire ne doit pas effacer celle qui l'a précédée, et qui a révélé la gravité des fêlures de notre société : celle des « gilets jaunes ». Dans ce contexte, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est un objet politique majeur. Acquis démocratique, il est le moment par excellence où doivent se confronter les attentes à l'égard du système social et les dispositions à même d'assurer son financement. Rappelons que l'enjeu est de taille : de l'ordre de 500 milliards d'euros. Il mérite que l'on s'y attarde un instant. C'est donc le moment de s'interroger sur la part de l'effort que les Français souhaitent consacrer à la santé, aux retraites, à la famille, au vieillissement. Cet effort est légitime ; rappelons que d'autres le sont tout autant : l'éducation et la formation professionnelle, mais aussi la culture ou la défense, pour n'en citer que quelques-uns. Aucun sujet n'est tabou, bien au contraire, mais les questions doivent être clairement posées. Or il semble à la commission des affaires sociales que ce projet de loi prend le plus grand soin à les éluder très largement. Sur la santé, le système public donne l'impression d'être hors de contrôle malgré les efforts budgétaires déployés. Les soignants fuient l'hôpital, certes épuisés par la crise, mais surtout en perte de sens dans des organisations qu'ils ne comprennent plus. Il est désormais certain que le Ségur de la santé n'y suffira pas, mais quel cap donner à présent au système de santé ? Sur l'autonomie, les années passent et nous rapprochent de plus en plus d'un véritable mur de financement, que les évolutions démographiques rendent inéluctable. Le diagnostic est clairement posé par les rapports qui s'empilent. Mais faute d'avoir répondu à la question cruciale du financement, la réforme s'est enlisée et le dossier patine. Qui doit assumer le financement de l'autonomie ? Les personnes concernées et, le cas échéant, leur patrimoine ? Les jeunes retraités pour préparer l'avenir ? La société dans son ensemble, mais, dans ce cas, sous quelle forme : l'impôt, l'assurance obligatoire ? Cette question relève-t-elle de l'aide sociale pour les plus pauvres ou d'une assurance généralisée ? Le système actuel proclame la seconde, mais ne finance que la première, et encore partiellement. Aucune réponse n'ayant été apportée à ces questions, la branche autonomie reste une coquille vide qui ne fait que labelliser des dispositifs existants. Ce ne sont pas les dispositifs proposés par le PLFSS qui suffiront à répondre aux enjeux. Sur les retraites, faut-il rappeler que les paramètres sont bien identifiés entre le niveau de vie que l'on souhaite garantir aux retraités et les efforts que l'on est prêt à consentir pour y parvenir ? Là encore, notre système doit s'adapter à des évolutions démographiques. La France vieillit : il faut faire en sorte qu'elle puisse en assumer les conséquences pour des générations moins nombreuses et confrontées de surcroît à des conditions économiques difficiles. La réforme des retraites la plus astucieuse et la plus complexe ne fera pas disparaître ces paramètres qui s'imposent à nous. Comme les années précédentes, la commission invite le Sénat à prendre ses responsabilités, sans tarder davantage et sans bercer les Français de contes qui ne dureront que le temps d'une campagne présidentielle. Ils ne sont pas des enfants et n'ont pas manqué de le faire savoir. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale devrait donc être l'occasion d'aborder ces grands enjeux et de se projeter dans l'avenir. Au lieu de cela, que nous propose ce texte ? Rien sur l'avenir, en tout cas, puisque la trajectoire pluriannuelle ne porte aucune trace d'action volontariste. Elle ne se fait en quelque sorte que le sismographe des effets de la croissance envisagée sur les comptes sociaux. Pour les décisions, il est acté qu'il en faudra, mais elles viendront plus tard. Nous pensons qu'une telle position n'est pas tenable et nous vous proposerons d'en tirer les conséquences. Pas grand-chose non plus sur la santé : le projet de loi de financement s'est mué cette année en catalogue de mesures éparses qui auraient souvent mieux trouvé leur place ailleurs. Entre l'encadrement des mesures de contention en psychiatrie, dont on peinera à nous expliquer pourquoi, après deux censures du Conseil constitutionnel, elles n'ont pu faire l'objet d'un texte spécifique, ou les aménagements par petites touches de la répartition des compétences entre les différentes professions de santé, on hésite, malgré le sérieux des sujets, entre l'inventaire à la Prévert et la complainte du progrès Pour redonner sa portée au PLFSS, la commission des affaires sociales a pris le parti de le recentrer sur sa vocation première, telle que la Constitution la définit, c'est-à-dire les questions de financement, qui à nos yeux se posent de façon cruciale cette année encore. Elle vous propose donc de supprimer toute une série de dispositions qui n'ont pas leur place dans ce texte et appelle à une saisine du Conseil constitutionnel sur ce point, afin qu'il structure clairement sa jurisprudence. Elle a de ce fait appliqué avec rigueur, me semble-t-il, les irrecevabilités spécifiques qui s'y attachent. L'enjeu est celui de la démocratie : les délais constitutionnels ne doivent pas forcer la main des parlementaires pour examiner à la va-vite diverses mesures d'ordre social qui seraient la « voiture-balai » du quinquennat Le PLFSS n'est pas le succédané d'une loi Grand Âge ayant renoncé à ses ambitions ou d'une loi Santé qui en serait dépourvue. C'est donc dans cet état d'esprit que nous abordons l'examen de ce texte, avec des objectifs clairs il ne suffit pas de se gargariser de l'excellence de notre modèle social ; encore faut-il lui donner les moyens de se renouveler et de s'adapter afin que nous puissions en faire non pas une parenthèse dans l'histoire, mais bien un legs pour les générations futures. Nous passons

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, face à la crise sanitaire qui a ébranlé le pays et mis en tension notre système de santé, et singulièrement les services hospitaliers, le Gouvernement a enfin choisi de ne pas poursuivre les réductions de dépenses pour l'hôpital. Après quatre ans de coupes claires, soit plus de 4 milliards d'euros depuis 2017, vous maintenez, monsieur le ministre, le même niveau- hors Ségur -que l'année dernière. Cette pause est la bienvenue, mais va-t-elle suffire à redresser la barre ? Les personnels sont épuisés et leurs conditions de travail ne leur permettent plus d'assurer leur mission dans de bonnes conditions, ce qui ne peut que nuire à la qualité des soins. Outre la nécessité de dégager des moyens suffisants, il s'agit de les rendre pérennes, ce que vous n'êtes visiblement pas prêts à faire. L'Ondam, sacro-saint objectif que nous n'avions jamais pu faire évoluer malgré les mobilisations syndicales et politiques, a dépassé fort heureusement la barre des 9 % d'augmentation en 2020, et le pouvoir à l'hôpital a quelque peu échappé aux technocrates pour laisser les équipes s'organiser, s'entraider au mieux des intérêts des patients. Mais pour 2022, retour à un Ondam inférieur à l'augmentation du coût des dépenses de santé, qui se situe entre 4 % et 5 %. Vous ne tirez donc aucune leçon de ce que nous sommes en train de vivre. Le Gouvernement semble pressé d'en finir avec la crise sanitaire pour reprendre sa politique là où il l'avait laissée, c'est-à-dire en réduisant et en contraignant encore et toujours les budgets. Ce budget, présenté comme exceptionnel par le Premier ministre, est en réalité une poursuite de l'offensive contre notre système de sécurité sociale. Après avoir décidé en 2020 de faire payer à la sécurité sociale la crise sanitaire et ses conséquences économiques, le Gouvernement poursuit sa logique de fiscalisation de la sécurité sociale. Nous sommes passés en quinze ans d'un financement de l'assurance maladie majoritairement par les cotisations sociales à un financement aux deux tiers par la CSG et les taxes. En réalité, les assurés sociaux perdent 75 milliards d'euros en exonérations de cotisations sociales et paient 75 milliards d'euros en TVA et en CSG pour compenser les pertes. Faire les poches des assurés sociaux, des retraités, sans parler de l'obligation d'avoir recours à des mutuelles ou à des assurances pour être mieux remboursé : on est loin du « 100 % sécu », qui a pourtant fait ses preuves pendant la pandémie ! On est loin de la sécurité sociale universelle, contrairement au discours du Gouvernement sur sa « grande sécu Nous refusons cette fiscalisation de la sécurité sociale, qui conduit à une mainmise de l'État- et, surtout, de Bercy -sur elle, qui traque tout ce qui est dépenses sociales. La sécurité sociale est confrontée à une crise de financement entretenue par les multiples exonérations de cotisations sociales qui viennent assécher ses ressources, d'autant que toutes ne sont pas compensées. Le Gouvernement reste fixé sur les dépenses, pensant s'en sortir par une reprise de l'activité économique, ce qui est parfaitement illusoire. Les exonérations de cotisations, qui ont doublé depuis 2013, se poursuivent. En conséquence, les recettes de la branche maladie restent inférieures à leur niveau de 2018, alors que cette branche est soumise à une augmentation des dépenses sans précédent avec la pandémie. Un petit rappel s'impose : l'ensemble des niches sociales s'élève à 90 milliards d'euros. Ces choix politiques assumés ont de violentes conséquences sur notre système de santé puisqu'en 2022, il manquera 21 milliards d'euros pour financer les dépenses de santé, soit l'équivalent de l'allégement lié au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Le fameux « trou de la sécu », qui est totalement organisé, est utilisé par le Gouvernement pour justifier les régressions sociales. Plutôt que d'assumer le coût de la crise sanitaire en empruntant à un taux négatif, comme l'État le fait actuellement, vous avez préféré laisser l'ardoise à la sécurité sociale pour faire payer la pandémie par les cotisations des assurés sociaux. Fidèles aux valeurs et aux principes qui ont permis l'édification de la sécurité sociale dans notre pays, nous sommes pour la suppression des exonérations de cotisations sociales et favorables à un retour de l'autonomie du budget de la sécurité sociale vis-à-vis de l'État, ainsi qu'à sa gestion par des administrateurs élus par les salariés et leurs ayants et leurs ayants droit. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, en prévoyant de faire financer la perte d'autonomie sur le dos des salariés et des retraités, porte atteinte au principe de partage de la valeur créée, qui fonde notre système de protection sociale. La crise sanitaire sans précédent qui a secoué notre pays, comme l'ensemble du monde, et qui n'est pas terminée, a mis en évidence comme jamais les failles de notre système de santé, creusées par les choix politiques faits depuis vingt ans. L'hôpital a tenu le coup grâce à l'engagement des personnels, mais à quel prix ? Celui d'un épuisement généralisé et d'une exigence partagée d'un changement de politique à leur égard. Or, après qu'ils ont été envoyés au front sans protection, après qu'ils ont été applaudis le soir à vingt heures, leurs conditions de travail ne cessent de se dégrader. De plus, on a assisté à une stigmatisation des personnels, accusés de ne pas se faire vacciner suffisamment vite. Une défiance telle s'est propagée que des contrôles de leurs arrêts de travail ont été organisés, et certains personnels ont même perdu leur emploi faute de vaccination. Je défends, comme l'ensemble de mon groupe, la vaccination, mais il y avait d'autres mesures à prendre que cette entorse sans précédent au code du travail, comme si l'on pouvait se passer d'elles et d'eux pour faire tourner les services, alors que la pénurie de personnel se fait sentir partout. La colère, l'amertume sont palpables dans tous les services. Selon une étude parue au printemps dernier, si c'était à refaire, trois médecins sur dix choisiraient une autre profession. Toutes les professions médicales et paramédicales sont touchées. Les contreparties financières à leur engagement dans la crise sanitaire dégagées par le Ségur de la santé sont jugées insuffisantes, car elles représentent en réalité un rattrapage de dix ans de blocage des salaires. Et il a fallu des réajustements, car beaucoup de catégories professionnelles, notamment dans le secteur médico-social, avaient été oubliées et le sont encore aujourd'hui. Vous nous dites, monsieur le ministre, que si des lits sont fermés- 13 300 depuis 2017, dont 5 700 en pleine crise sanitaire, et je ne fais pas référence à l'alerte récente du professeur Delfraissy -, c'est par manque de personnel. Mais seulement 15 000 recrutements sont prévus par le Ségur de la santé, soit en réalité 7 500 selon Bercy, ce qui fait à peine six postes par hôpital, quand les postes vacants représentent près de 20 % des effectifs. Pourtant, en un an, le nombre de départs d'infirmières et d'infirmiers exerçant dans le public a bondi de 43 %.

Face aux difficultés de recrutement dans les professions paramédicales et médicales, le Gouvernement fait comme si la crise sanitaire était l'unique cause de l'épuisement des professionnels de santé. Mais c'est oublier que si les moyens financiers avaient été débloqués en 2019 lors du plan Ma santé 2022 pour augmenter la capacité de formation des médecins et autres spécialités de santé, nous aurions pu, d'ici cinq ans, inverser la courbe de réduction du nombre des médecins généralistes pour 1 000 habitants. Ce n'est pourtant pas une crise de vocations, puisque, du côté des jeunes, l'élan pour les métiers de soins est toujours présent. Nous sommes certes passés d'un national à un fixé selon les capacités d'accueil des universités, mais les chiffres restent très bas compte tenu du manque de moyens Selon le sociologue de la santé Frédéric Pierru, les rémunérations ne figurent pas en tête des facteurs de satisfaction au travail : les soignants privilégient le soutien des collègues, des supérieurs, la reconnaissance du travail effectué et, bien entendu, les conditions de travail, qui déterminent la qualité de l'ambiance au sein des équipes. Rien n'est prévu dans ce PLFSS 2022 pour répondre à ces justes revendications. L'adaptation de la société au vieillissement, la nécessité de recouvrer notre souveraineté sanitaire avec une production de médicaments et de produits de santé en France, comme nous vous y invitons à travers notre proposition de loi portant création d'un pôle public du médicament et des produits médicaux, la mise en oeuvre d'une démocratie sanitaire qui accorde enfin une place aux personnels, aux usagers et aux élus locaux, une psychiatrie digne du XXIsiècle : voilà des sujets urgents à traiter. Ce PLFSS est un empilement d'articles qui ne font ni sens ni cohérence. Le monde a changé, l'hôpital public doit redevenir la place forte d'un nouveau modèle de santé. Il est essentiel, par exemple, de créer toutes les conditions d'une coopération entre médecine de ville et médecine hospitalière, à l'heure où les déserts médicaux étendent leur spectre sur l'ensemble du territoire. Il est plus que jamais indispensable d'avoir une vision à long terme. Or cette vision à long terme, cette impulsion, c'est à l'État de la donner. Hélas ! monsieur le ministre, c'est tout le contraire que vous faites. Vous lancez des appels à projets auprès des ARS et vous attendez leur retour pour faire vos choix. Mais ce n'est pas ce qu'on attend d'une politique de santé nationale ! Sans vision globale, c'est la déliquescence généralisée. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe CRCE a décidé de déposer cette motion tendant à opposer la question préalable. Et j'espère qu'elle sera votée ! Personne ne demande

Dans les hôpitaux, en médecine de ville, dans les ministères et dans les agences régionales de santé, je défends les fonctionnaires ! Par ailleurs, vous avez déploré que la sécurité sociale soit en partie financée par la CSG.

Le scrutin est ouvert.

après sept années passées comme rapporteur général de la commission des affaires sociales, je mesure pleinement la charge qui vous revient. Nous savons tous ici pouvoir compter sur vos compétences et sur la sagesse de vos analyses pour éclairer notre assemblée et convaincre, je l'espère, le Gouvernement

par l'exécutif. Je pense notamment à un sujet majeur, la non-compensation des exonérations et suppressions de cotisations, décidée au mépris de la loi Veil de 1994 et à rebours des dispositions organiques.

lui-même. Ministres ou rapporteurs, chacun est dans son rôle. Pour les uns, le verre est à moitié plein ; pour les autres, il est à moitié vide.

le présent texte donne-t-il un cap ? Oui, si l'on considère les efforts consentis pour les revalorisations des salaires des soignants dans de nombreux secteurs ; pour l'amélioration des droits sociaux des travailleurs indépendants et pour le développement de la téléconsultation ; pour le versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne et, plus généralement, la mise en place progressive du modèle domiciliaire pour les personnes dépendantes, notamment avec l'augmentation tarifaire minimale et la transformation des Ehpad en centres de ressources.

le Gouvernement reste particulièrement flou quant à la gouvernance de cette cinquième branche, dont les enjeux sont non seulement financiers, mais aussi humains. La proximité qu'apportent les départements nous paraît vitale pour permettre aux personnes en perte d'autonomie de vivre à domicile le plus longtemps possible. Une question plus vaste encore nous taraude : celle du retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Avec le covid et le rattrapage salarial, le « trou de la sécu » se creuse à nouveau. Il nous appartient de remédier à cette situation, par souci de responsabilité à l'égard des assurés et des Français dans leur ensemble. Pourtant,

Espérons d'ailleurs que les reports temporaires liés au covid seront honorés en 2022 et qu'ils ne creuseront pas plus le déficit. Attardons-nous un instant sur les fraudes. Je regrette qu'un seul et unique article reprenne les mesures de la proposition de loi votée au Sénat en 2020 et que les trois principales caisses ne livrent leurs estimations de la fraude qu'après l'examen du PLFSS. Réjouissons-nous quand même

En matière d'économies, évoquons aussi la pertinence des soins, dont vous nous dites qu'elle monte en puissance. Je note bien quelques mesures ou intentions ponctuelles, mais je constate surtout l'absence de vision stratégique, que je signalais déjà dans le rapport de la mission face à cet enjeu majeur- rappelons que 20 % à 30 % des actes sont inutiles ou redondants -, les réponses sont trop timides. Le dossier médical

c'est celle de l'équilibre. Elle n'est pas à l'ordre du jour, répond le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux. J'approuve tout à fait ce point de vue, qui n'empêche pas pour autant de réfléchir au retour à l'équilibre de ce régime à moyen terme. Le rapport Tirole-Blanchard, relatif aux finances publiques, mérite en ce sens toute notre attention. Plutôt qu'un âge de départ à 64, 65 ou 67 ans, il retient une « fenêtre de départ

Rappelons que l'âge réel de départ à la retraite est déjà proche de 63 ans, que la durée de cotisation est de 42,6 ans aujourd'hui

jusqu'en 2004, les médecins généralistes avaient une obligation de garde. Aujourd'hui, seuls 39 % d'entre eux y participent. Il faut donc revoir l'organisation de la garde par les médecins de ville afin d'éviter la thrombose des urgences hospitalières.

aussi à moins de six mois de l'élection présidentielle. La première leçon que nous retiendrons du covid, c'est la place de la santé dans la hiérarchie des valeurs de notre société. Alors que nous glissions sur la pente de plus en plus financiarisée d'une société high-tech et numérique, nous avons brutalement pris conscience que la santé- la vie, tout simplement -était bien l'essentiel. Sans elle, il n'y a plus de société, les robots ne nous ayant pas encore tous remplacés et éliminés de la planète. Cette réaction pour notre survie, quoi qu'elle en coûte, a été globalement partagée par nos concitoyens, même si les modalités de protection collective ont pu être débattues et sont encore discutées : la prolongation du passe sanitaire

Je pense au maintien de la présence en milieu scolaire comme à l'exceptionnel soutien à notre économie, qui permet, aujourd'hui, un premier redressement de la trajectoire des comptes sociaux que nous avons à examiner. Dans un contexte de précampagne présidentielle, où les propositions d'extrême rigueur des uns le disputent à la plus grande démagogie des autres, je salue le double signal que constituent le redressement de la trajectoire des comptes et l'effort de dépenses raisonnable pour la santé. Il nous revient de veiller au financement des prestations d'aujourd'hui, afin qu'elles ne pèsent pas de manière déraisonnable sur les générations futures. Le régime général était redevenu excédentaire en 2018. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoyait même un quasi-retour à l'équilibre du régime général et du fonds de solidarité vieillesse d'ici à 2023. La crise est venue durablement bouleverser ces prévisions, avec un effort de près de 35 milliards d'euros en 2020 et un déficit attendu de 15 milliards d'euros à l'horizon 2024-2025. Nous le savons tous : les dépenses de santé, dans toute l'acception du terme- bien-être physique, psychique et social -, continueront de croître, parce que nous vivons de plus en plus longtemps et que nombre de soins accompagnent cette augmentation de l'espérance de vie. La prévention et les bonnes règles d'hygiène de vie ne sont ni suffisantes ni suffisamment partagées. surcroît, les soins auxquels nous pouvons avoir accès sont de plus en plus sophistiqués et onéreux. Les progrès de la médecine, auxquels nous aspirons tous, ont un coût. Ils impliquent des thérapies chères.

effort ne saurait nous exonérer d'une extrême vigilance quant à l'évolution des comptes sociaux. La maîtrise de ces dépenses passe autant par la place effective que doivent retrouver les élus dans les décisions de proximité que par nos amendements au PLFSS. Les élus ont été exclus des prises de décision. Ils sont cantonnés dans un rôle de bienveillante surveillance. Les pleins pouvoirs ont été donnés à l'administration hospitalière et de santé.

113 en 2023, 127,9 en 2024 et 143,2 en 2025, il faudra bien s'interroger sur le financement. Pouvons-nous

proviennent des revenus d'activité, au moment même où l'on nous annonce des revenus financiers atteignant des niveaux inégalés : les récents records du CAC 40 en attestent. Si l'on veut diminuer les charges des entreprises, réduisons les prélèvements sociaux afin d'alléger le coût du travail et d'augmenter, en même temps, les revenus de ceux qui fournissent ce travail. Le Gouvernement l'a fait en 2018, en décidant une baisse des cotisations sociales supérieure à la hausse de la CSG. Cette mesure a permis une progression du pouvoir d'achat des actifs. actifs. En 2018 et 2019, la transformation du CICE en une réduction de six points de cotisations maladie suivait la même logique. Tout ce qui a pour effet de réduire les prélèvements sociaux sur le travail

De même, le taux de CSG sur les revenus d'activité est égal au taux applicable aux revenus du patrimoine et aux produits de placement : un allégement des prélèvements sur les revenus d'activité permettrait une meilleure reconnaissance du travail.

Les retraités ont souvent acquis leur propriété, alors que de nombreux actifs sont encore en voie d'accession et apportent toujours un soutien financier à leurs enfants, étudiants pour certains. Tout en épargnant les petites retraites, bien sûr, il ne serait pas injuste de demander un effort aux premiers bénéficiaires. Parallèlement, le ticket modérateur, qui ne modère pas les complémentaires, doit être repensé au terme d'une réflexion approfondie sur la « grande sécu » et la place des mutuelles.

notamment immédiate la perception des aides applicables au secteur des services à la personne, lequel va nécessairement croître dans les années à venir, avec l'allongement de l'espérance de vie. Il est aussi prévu d'assouplir les régimes de déclaration pour les travailleurs indépendants : il s'agit là d'une mesure bienvenue pour ces professionnels, frappés de plein fouet par la crise sanitaire.

Je salue également la prise en charge dans le droit commun de la télésurveillance par l'assurance maladie, tout comme la poursuite de l'évolution, engagée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, au regard des médicaments faisant l'objet d'autorisations temporaires

tarif plancher national de 22 euros de l'heure pour les services à domicile et étend les missions des Ehpad à une offre d'accompagnement à domicile des personnes en perte d'autonomie.

Le Gouvernement nous promet une sécurité sociale structurellement déficitaire, aussi loin que courent ses tableaux prévisionnels. Or, maintenir la sécurité sociale en déficit sans perspective, c'est envoyer à la Nation un message politique : celui d'une protection sociale qui serait trop onéreuse, au-dessus de nos moyens. C'est aussi adresser à celles et ceux qui travaillent dans les domaines de la santé et du médico-social le message que ces activités pèsent sur le pays, alors même qu'elles en sont l'une des principales richesses, qu'elles constituent un bien précieux : celui de la solidarité nationale. Ce fut l'honneur de la gauche d'avoir presque rétabli les comptes sociaux, même si ce fut une erreur de n'avoir pas préservé nos hôpitaux de cet effort.

Nous n'esquiverons pas non plus le débat sur l'autonomie. En approuvant la création de la cinquième branche, nous avons- peut-être par excès de respect pour la parole du Gouvernement -accepté que le cadre en soit posé ultérieurement, lors de l'étude d'un projet de loi sur l'autonomie et la dépendance. Las, la parole n'a pas été tenue. Le Gouvernement sature l'agenda du Parlement de textes opportunistes et souvent bâclés et refuse d'affronter ce qui est, de fait, la grande question irrésolue de notre protection sociale. Vous faites naître la cinquième branche également en déficit- déficit de cadrage, de vision, de dispositifs, et déficit financier. Ma collègue Michelle Meunier y reviendra. Les retraites sont la seconde esquive de ce budget. La grande réforme systémique s'est perdue dans un agenda plus que jamais livré aux derniers calculs du Président, tandis qu'est lancé le grand concours de la surenchère du report de l'âge légal. L'esquive consiste ici à ne pas dire aux Français que l'on projette d'ajouter encore des conditions nouvelles à l'obtention d'une pension complète, alors même qu'ils sont de plus en plus nombreux à ne plus être en activité à l'heure du départ, et que la dégradation des conditions de travail rend cette perspective socialement injuste et souvent physiquement irréaliste Enfin, notre système de santé est l'objet de la troisième esquive. Vous connaissez évidemment, monsieur le ministre des solidarités et de la santé, la gravité de la situation de notre système de soins. Vous savez, bien sûr, que nos hôpitaux publics sont en voie d'affaissement- d'effondrement, même, selon certains.

Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, continuer à arguer des revalorisations- certes bienvenues -du Ségur de la santé pour affirmer que vos décisions sont à la hauteur de la crise hospitalière. Chaque jour apporte un démenti par les départs de soignants, par les fermetures de lits, et par la reprise, dès le sortir de la première vague, d'une logique administrative qui étouffe les soignants et dégrade l'attractivité des métiers de l'hôpital. Un hôpital n'est ni une administration ni une entreprise. Épuisés par ces deux logiques, ce sont les soignants qui s'en vont. Pour ce qui est des soins de ville,

Que des évolutions soient nécessaires, nous vous l'accordons. Cependant, elles doivent être effectuées dans le respect des temps : d'abord, le temps des discussions dans le cadre des conventions, puis l'intervention de l'exécutif et du Parlement si les intérêts et les besoins de la population sont insuffisamment respectés. Or vous faites tout le contraire : après avoir écarté la négociation conventionnelle, vous écartez les syndicats professionnels et vous imposez des décisions qui braquent les uns ou les autres, et qui produisent, je vous en avertis, un malaise qui finira par se muer en des renoncements professionnels.

Il nous faut partir des besoins des territoires, et ensuite- ensuite seulement -procéder aux arbitrages budgétaires qui demeurent, bien sûr, indispensables. L'outil de régulation que constitue l'Ondam montre en ce sens ses limites. La maîtrise qu'il porte s'impose avant toute délibération sur les besoins en matière dans nos territoires comme au Parlement où aucun débat sur les besoins sociaux de la Nation n'a lieu en amont de la délibération budgétaire. Nous pensons qu'il est temps de changer de paradigme sur cette question. L'Ondam est l'outil dépassé d'une époque passée. Vous l'avez compris, nous ne pouvons nous satisfaire de ce PLFSS. Le Parlement doit être à même de mieux déterminer les besoins de la Nation en matière de santé, dans un cadre démocratique. Ne passons pas à côté de cette tâche, à un moment où les acteurs de santé, les élus locaux et nos concitoyens demandent à être associés à ces choix fondamentaux pour notre collectivité nationale. La sécurité sociale a su tenir la société au moment de la crise, et nous avons été reconnaissants de bénéficier d'un tel système. Nous avons trouvé un consensus dans nos rangs sur l'aspect essentiel de l'ensemble des métiers et des dispositifs qui nous ont permis de faire face à l'épidémie. Nous devons maintenant

au regard des nombreux enjeux qu'il recouvre et de son importance pour le quotidien des Français. Il l'est d'autant plus cette année. Il l'est au regard du calendrier politique dans lequel il s'inscrit, puisqu'il s'agit du dernier PLFSS du quinquennat. Il l'est également de par le contexte sanitaire inédit. La pandémie qui a frappé le monde, qui nous a frappés, a exigé des réponses fortes et immédiates de la part du Gouvernement, afin de protéger les Français.

Ce budget de la sécurité sociale confirme, en premier lieu, les engagements du Ségur de la santé en matière de revalorisations salariales, d'une ampleur inédite pour l'ensemble des secteurs. Ainsi, 2,7 milliards d'euros de dépenses supplémentaires sont prévus en 2022, portant le total des revalorisations à plus de 10 milliards d'euros. Ce budget comprend également des mesures nouvelles au profit des salaires les moins élevés des praticiens hospitaliers ou encore des sages-femmes, dont le rôle au sein de notre système de santé est essentiel. Il confirme donc, comme je viens de le rappeler, les engagements pris, mais il consacre également de nouveaux droits pour répondre aux besoins des Français. Je pense à la possibilité de se faire prescrire des lunettes chez un orthoptiste- alors que nous savons que le délai moyen d'attente chez un ophtalmologue s'élève à six mois

2,8 millions de Français seront concernés par ce dispositif, dont le caractère protecteur est renforcé par ce budget. La généralisation du recours à l'intermédiation financière des pensions alimentaires compensera

En aucun cas l'enfant, dont l'intérêt supérieur doit toujours primer, ne doit être la victime collatérale d'une séparation ou d'un divorce. Je pense, enfin, au remboursement intégral de la contraception pour les 3 millions de femmes de moins de 26 ans. Il s'agit d'une mesure forte, d'autant que plusieurs études montrent que l'achat de moyens de contraception est davantage effectué par les femmes. Une réflexion devra d'ailleurs être engagée être engagée sur les disparités qui subsistent entre les femmes et les hommes en matière de connaissance des dispositifs existants, et sur la nécessité de mieux responsabiliser les hommes sur la contraception afin de parvenir à une réelle égalité en la matière.

3,5 milliards d'euros, dont 2,8 milliards d'euros de revalorisations salariales, 250 millions d'euros pour les services à domicile, 70 millions d'euros pour pour la médicalisation et la modernisation des Ehpad et 450 millions d'euros pour l'investissement. Il s'agit donc d'un budget considérable, à la hauteur des enjeux auxquels cette branche devra faire face. Nous savons combien la perte d'autonomie d'un parent ou d'un grand-parent peut être source d'inquiétude pour la famille et implique des aménagements importants pour subvenir à ses besoins. Il nous faut donc renforcer la qualité de l'offre à domicile tout en poursuivant nos investissements à destination des Ehpad et de leur modernisation. L'article 30 du PLFSS, relatif à la réforme et à la revalorisation de l'offre de services à domicile en matière d'autonomie, répondra à cet objectif en faisant évoluer les services de soins infirmiers à domicile afin de prendre davantage en compte les besoins en soins des personnes par rapport à leur degré d'autonomie. La nouvelle mission de centre de ressources territorial pour les Ehpad, créée à l'article 31 de ce PLFSS, apportera un appui aux professionnels du territoire, notamment la mise à disposition d'expertise gériatrique, ainsi qu'un accompagnement renforcé pour les personnes âgées en perte d'autonomie nécessitant un accompagnement à domicile intensif. Enfin, nous nous félicitons des apports de l'Assemblée nationale visant à renforcer le congé du proche aidant, en élargissant le champ du bénéficiaire de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) aux proches aidants de personnes dont le handicap ou la perte d'autonomie peuvent nécessiter une aide régulière. La revalorisation au niveau du SMIC du montant de l'allocation journalière était attendue, et légitime au vu de l'engagement de ces personnes. En tout état de cause, le groupe RDPI salue et soutient pleinement les orientations de ce budget. d'un budget à la hauteur des attentes, qui consacre de belles avancées sociales à destination de tous les Français- en particulier de ceux qui en ont le plus besoin : nos aînés, les personnes en situation de handicap, ainsi que celles et ceux qui leur viennent en aide Ce budget est également à la hauteur des enjeux auxquels notre pays fait face. Je pense en particulier au secteur hospitalier, aux femmes et aux hommes dont la pandémie mondiale a révélé une fois de plus le rôle central, crucial pour notre pays et nos concitoyens. La parole

la fois les effets à long terme de la crise sanitaire sur les comptes sociaux et le souhait de nous tourner vers l'avenir, est susceptible de renforcer l'accès à la santé pour l'ensemble des Français. Les comptes sociaux

d'euros en 2021. Ce déficit est essentiellement supporté par la branche maladie, victime d'un effet de ciseau entre la contraction des recettes et la hausse des dépenses liées aux mesures du Ségur de la santé et à l'amortissement des effets de la crise.

Ces hypothèses se fondent sur une amélioration durable de la situation sanitaire, appuyée sur la poursuite de la campagne vaccinale, une vigilance renouvelée en matière de prévention des contaminations et un suivi actif de l'évolution des formes du virus. Si 88 % de la population majeure est désormais vaccinée- c'est un succès -, la pandémie n'est pas encore vaincue. Elle regagne du terrain en France comme dans le monde et nous devons rester pleinement Nous débattrons de plusieurs questions importantes allant de l'organisation de notre système de soins à la réforme des retraites- sans oublier la question du grand âge, essentielle à mes yeux. J'aimerais, pour commencer, saluer les avancées apportées par le texte pour renforcer l'accès aux soins et aux droits sociaux. Les revalorisations salariales des soignants et du secteur médico-social se poursuivent, en accord avec les conclusions du Ségur de la santé. À ce sujet, il serait souhaitable, monsieur le ministre, de renforcer la lisibilité des mesures de revalorisation successives adoptées afin de mieux identifier les catégories de personnels qui ne bénéficient pas encore du complément de traitement indiciaire de 183 euros net par mois. Ces « oubliés du Ségur » subissent de

les plus vulnérables. souffre d'une répartition inégale des professionnels sur le territoire et d'un fort cloisonnement, justifiant un élargissement progressif, depuis 2016, du pouvoir de prescription des orthoptistes. Je suis favorable à cette tendance, tout en estimant nécessaire de préserver le lien entre patients et médecins ophtalmologues pour certains contrôles oculaires. favorable à la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 26 ans, mais suggère de l'étendre aux hommes de la même tranche d'âge. Le remboursement des préservatifs masculins permettrait de prévenir les risques de transmission des infections sexuellement transmissibles (IST) et de grossesses non désirées.

financière pour faciliter le versement des pensions alimentaires, sachant que le taux d'impayé se situe autour de 30 %. Il s'agit d'une évolution majeure pour lutter contre la pauvreté des familles monoparentales, souvent constituées de mères célibataires. Nous devons en outre réfléchir,

que l'accès facilité aux médicaments innovants sont également des mesures bienvenues. La retraite à mille euros pour les exploitants, la suppression de la surcotisation sur la prime de feu des sapeurs-pompiers et la délivrance de substituts nicotiniques par le pharmacien constituent aussi des avancées. Le Gouvernement s'est engagé à présenter un amendement pour compléter le dispositif de la proposition de loi présentée présentée par Paul Christophe et adoptée par le Sénat la semaine dernière. En revanche, nous devons aller plus loin pour lutter contre les déserts médicaux, en particulier pour renforcer l'accès aux soins psychiatriques et aux médecins généralistes. Je présenterai des amendements visant à instaurer un conventionnement sélectif dans les zones surdotées. Je regrette que les amendements que j'avais déposés tendant à obliger les jeunes médecins généralistes

ans au seul renforcement des effectifs de soignants, soit cinq soignants supplémentaires en moyenne par Ehpad. Nous passerions ainsi à un encadrement de 0,6 à 0,7 équivalent plein (ETP) par pensionnaire. Cette mesure est demandée depuis des années par les directeurs, le personnel et les familles. Si nous pouvons comprendre l'étalement dans le temps de ces créations d'emploi en raison de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas comprendre le renoncement au renforcement des effectifs en Ehpad,

l'avenir des seniors, d'autant que 2,5 millions de personnes seront en perte d'autonomie en 2050, soit deux fois plus qu'en 2015. Je suis favorable à l'ouverture des Ehpad vers l'extérieur,

de nos concitoyens. La population française est vieillissante. Cette réalité implique un véritable questionnement sur le système de retraite. Si nous ne voulons pas pénaliser les retraités par une baisse du montant des retraites ni le niveau de vie des actifs par une augmentation des cotisations, le report

l'âge de la retraite à 64 ans. En complément de cette mesure paramétrique, nous devons favoriser la durabilité de l'emploi des seniors par l'action de trois leviers : la prévention, la formation continue et la transmission des compétences par le tutorat et le mentorat- Monsieur le ministre, si nous saluons l'augmentation des salaires des soignants- qui doit être équitable pour tous les intervenants -et les avancées apportées par le texte, nous déplorons l'absence de proposition d'une trajectoire financière pour une prise en charge décente de nos aînés, à domicile comme en établissement. La

Bien sûr, les comptes sociaux sont encore très marqués par la crise sanitaire, mais dans ce dernier PLFSS vous n'envisagez aucun choix budgétaire, aucune réforme structurelle pour retrouver l'équilibre. De surcroît, les réformes plus délicates à mettre en oeuvre comme la réforme des retraites ou la loi Grand Âge et autonomie sont reportées aux calendes grecques. Les familles sont les grandes perdantes de ce budget. En matière de politique familiale, les PLFSS se succèdent et se ressemblent. Le détricotage de notre politique familiale continue. Une fois de plus, la branche famille ne fait l'objet que d'un très petit nombre de mesures dans le PLFSS. Même si nous soutenons l'allongement du congé paternité pour les collaborateurs de professions libérales ou encore l'amélioration du recouvrement des pensions en cas de divorce, force est de constater que ces mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Cette absence est d'autant plus regrettable que la branche famille est excédentaire. Je rappelle que la bonne situation financière de cette branche s'est faite au prix d'importantes mesures d'économies qui ont affecté directement le budget des familles. Il s'agit de la modulation des allocations familiales, de la suppression du complément de libre choix d'activité majoré, ou encore de la modulation de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. Toutes ces réformes ne datent pas de 2017, je vous l'accorde, certaines ayant été introduites bien avant, en 2014. Cependant, votre gouvernement, monsieur le ministre, n'a pas fait le choix de revenir sur ces mesures- bien au contraire, puisque vous avez sous-revalorisé les prestations familiales en 2019. L'accumulation de toutes ces mesures fait perdre à la branche famille son rôle essentiel de compensation des charges de famille. Pourtant, la politique familiale constitue un investissement pour l'avenir. Enfin, il n'est pas légitime que les dépenses directement liées à l'épidémie de covid-19 soient assumées par la branche famille, et non par la branche maladie.

Actuellement, 18 % de la population vit dans un territoire qualifié de « zone sous-dense ». Cette raréfaction de l'offre de soins s'observe alors même que les besoins médicaux de la population s'intensifient en raison du vieillissement, de l'augmentation des maladies chroniques et de la croissance de la population. Monsieur le ministre, vous avez annoncé la fin des déserts médicaux d'ici cinq ans. Je m'étonne donc que ce projet de loi ne comporte aucune mesure financière pour lutter contre ces derniers et soutenir l'installation des médecins dans les zones sous-denses. Comment sortir de cette situation et offrir un accès aux soins équitable à l'ensemble de la population ? La télémédecine est une réponse limitée qui ne saurait pallier sur le long terme l'absence de médecins dans les déserts médicaux. La fin du aura sans doute des effets, mais seulement dans une dizaine d'années. Il n'est pas acceptable que, dans notre pays, certains territoires soient totalement dépourvus de professionnels de santé. Les Français qui rencontrent des difficultés d'accès aux soins n'en peuvent plus d'attendre Pendant l'examen du PLFSS, nous proposerons des mesures fortes pour combattre les déserts médicaux, notamment la création de zones franches médicales dont le périmètre sera défini par les ARS en concertation avec les élus des collectivités territoriales concernées. Si l'on veut une juste répartition de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national, il est nécessaire d'accompagner les médecins et d'associer les élus. Le droit à la santé, composante essentielle du pacte républicain, implique l'égal accès de chacun aux soins nécessités par son état de santé et justifie que l'État, garant de l'égalité et de la solidarité, se trouve en première ligne en matière de santé publique. La parole

dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale du mandat est aussi celui du bilan des cinq années écoulées. Ce PLFSS comporte plus d'avancées que les précédents, ... Ah ! ... mais est-il pour autant à la hauteur des enjeux et répare-t-il les logiques « austéritaires » des quatre précédents

Chacun a-t-il été assuré face aux risques ? Tout le monde a-t-il été invité, à la mesure de ses moyens, à participer aux charges ? Un premier constat s'impose quant aux 38 milliards d'euros exceptionnels que coûtera la covid-19. Quelles ressources exceptionnelles le Gouvernement a-t-il mobilisées les profits et distributions de dividendes tout aussi exceptionnels des grands groupes ou une contribution exceptionnelle des revenus des ménages les plus aisés qui ont enregistré des records d'épargne et d'augmentation de leurs patrimoines

Quant au Ségur de la santé, rattrapage partiel de longues années de décrochage salarial, il prévoit 10 milliards d'euros supplémentaires- désormais compris dans la base de l'Ondam et donc récurrents -que le retour à un taux de croissance de croisière ne pourra absorber. Quelles recettes nouvelles le Gouvernement mobilise-t-il Aucune ! Comment s'étonner en ce cas de retrouver l'équivalent de cette dépense représentant deux tiers, voire la totalité du déficit structurel des projections financières en 2025 ? Sans apport de nouvelles recettes,

Voilà le constat principal qui délégitime l'économie générale de ce budget- comme celle des budgets précédents. La protection sociale ne peut prospérer, ni même être défendue, quand les inégalités augmentent, quand un clan reste intouchable. Malgré cela, la sécurité sociale a joué son rôle d'amortisseur social, mais aussi économique, par le recours massif à l'activité partielle qui a permis de préserver une grande partie des emplois et des compétences. Grâce à cela, la relance a été rapide. La branche maladie et la branche autonomie ont engagé le rattrapage partiel d'années de déflation salariale,

recettes suffisantes. L'offre a été contrainte pour brider la demande, ce qui a aggravé les déserts médicaux, l'endettement de l'hôpital et l'effondrement de ses investissements. L'explosion des postes vacants dans tous les métiers- des aides-soignantes et infirmiers jusqu'aux médecins praticiens -a dégradé les conditions de travail et enclenché un cercle vicieux d'absentéisme, de démissions et de crise du recrutement. C'est alors que la crise sanitaire a percuté un système de santé dont vous aviez poursuivi la dégradation.

Par ailleurs, les 13 milliards d'euros dégagés pour désendetter l'hôpital ne doivent avoir qu'une finalité : lui permettre de se moderniser. Il ne s'agit pas de satisfaire aux injonctions de Maastricht et de réduire l'endettement des administrations publiques en bloquant leurs investissements. La réduction de l'endettement, lequel est dû à l'insuffisance des Ondam, doit améliorer l'autofinancement et le recours à l'emprunt sur des bases saines et pluriannuelles. L'État, enfin, doit tenir son engagement de reverser aux établissements de santé les crédits sous-exécutés. Il fallait donc un électrochoc. Vous présentez une loi de financement plus satisfaisante que vos budgets précédents, mais, à l'image de ce que vous prévoyez pour la branche autonomie, faute de dégager les ressources nécessaires dans le cadre d'une programmation pluriannuelle ambitieuse, le compte n'y est pas. De plus, la dette sociale conduira, élections passées, à de nouvelles baisses des dépenses. S'agissant des autres branches, la grande loi sociale du quinquennat, rebaptisée « Générations solidaires » à défaut d'être née, promise chaque année. Elle restera pourtant le rendez-vous social manqué du Gouvernement, lequel a préféré saturer le travail parlementaire de lois sécuritaires plutôt que de répondre à l'enjeu de la transition démographique à l'horizon de 2030. Dans cette transition aussi, la France prend du retard ! Si le projet de loi comprend des mesures positives, qui témoignent du virage domiciliaire, celles-ci

réduit ainsi les inégalités territoriales, ce qui va dans le bon sens, même si son aide sera d'autant plus importante que le département pratiquait un tarif bas,

Surtout, le tarif plancher non indexé demeure bien inférieur au tarif d'équilibre retenu il y a deux ans dans le rapport Libault. À défaut d'un changement radical de modèle économique, il installe durablement une sous-tarification des services. Nous soutiendrons pourtant des amendements concernant d'autres mesures de la branche autonomie. Là encore, une loi à la hauteur des enjeux nécessiterait d'importantes recettes nouvelles. Cela explique peut-être le recul du Gouvernement, lequel n'excelle que dans l'effort sur les dépenses. La branche AT-MP est, certes, à l'équilibre, mais reste curative et épuise en un quadrimestre son budget annuel de prévention.

L'iniquité des situations a entraîné des transferts de personnel de secteurs en situation de sous-effectif dramatique vers d'autres dont la situation relative s'améliorait. La pénurie s'est ainsi déplacée, sans que l'attractivité globale s'améliore, parce que les conditions de travail se dégradent En conclusion, le groupe écologiste soutient toutes les avancées, de la prise en charge de la contraception à la création des services autonomie, mais il faut construire la sécurité sociale des grandes transitions et lui allouer les ressources nécessaires. Ce projet de loi ne trace pas

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, dans la continuité de la motion défendue par ma collègue Laurence Cohen, je souhaite dénoncer les insuffisances et les dangers de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses propositions que Laurence Cohen vous a exposées- sans dogmatisme, monsieur le ministre ! Après dix-huit mois d'une crise sanitaire inédite, qui n'est pas encore arrivée à son terme, nous étions en droit d'attendre que le PLFSS pour

Chaque année, vous faites le choix de faire peser sur le budget de la sécurité sociale des mesures qui devraient être financées par le budget de l'État. Cela a concerné la crise des « gilets jaunes », puis celle du covid ; cette année, il s'agit des dépenses liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Nous avions déjà dénoncé l'an dernier cette méthode, qui aggrave le déficit de notre système de protection sociale. Malgré cela, la sécurité sociale a joué un rôle indispensable,

de l'article 40 est passée et a rendu irrecevables certains de nos amendements. Nous discuterons donc à la marge d'un texte dont les principaux arbitrages ne bougeront pas.

Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ! En limitant les recettes de la sécurité sociale, tout en lui faisant supporter le coût de la crise, vous creusez le déficit. En 2006, les cotisations sociales représentaient 50 % du financement de la branche assurance maladie, contre 34 % aujourd'hui. Au total, les exonérations de cotisations sociales représentent une perte de 75 milliards d'euros de recettes pour notre sécurité sociale. Imaginez ce que nous pourrions faire avec cet argent Depuis 2017, les économies infligées à l'assurance maladie représentent 18 milliards d'euros, dont 4,1 milliards sont à la seule charge des hôpitaux. Le bilan de cette politique, conjuguée au virage ambulatoire, est désastreux : 5 700 lits d'hospitalisation ont été fermés en 2020, en pleine crise sanitaire. Ces fermetures s'ajoutent aux 7 600 aux 7 600 lits déjà supprimés depuis 2017. De même, la France compte désormais moins de 3 000 hôpitaux et cliniques. Sous l'effet des réorganisations et des restructurations, vingt-cinq établissements ont fermé en 2020.

eux ont obtenu des revalorisations, bien insuffisantes, d'autres non. C'est juste assez pour essayer de diviser les professionnels entre eux. Vous avez cassé l'hôpital public à grands coups d'économies et de plans de retour à l'équilibre ; la crise du covid n'a été que le révélateur d'une gestion comptable appliquée à la santé depuis bien longtemps. Ce qui est vrai dans le soin l'est aussi dans la prise en charge de l'autonomie. On allait voir ce qu'on allait voir : enfin une grande réforme du grand âge et de l'autonomie ! Elle a fait « pschitt ! », disparue, envolée, tout juste recyclée dans quatre articles de ce texte. Ce n'est pas à la hauteur.

pour ces femmes qui vivent avec moins de 900 euros par mois, dans des conditions difficiles et avec une pénibilité qui brise les corps et les carrières. Vous vous êtes pourtant arrêtés au milieu du gué.

d'autres non, alors qu'elles exercent le même métier. Qui va payer pour que ces secteurs puissent garder leurs salariés ? Il manque aujourd'hui 250 000 aides à domicile, toutes structures confondues ; avec ces mesures, vous aggravez la situation. S'agissant de la réforme du financement de l'aide à domicile et de la création d'un tarif plancher, je tiens à rappeler que cette proposition avait été faite avec un minimum de 25 euros par mon prédécesseur Dominique Watrin et Jean-Marie Vanlerenberghe, dans un rapport de 2014 intitulé « L'aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer d'urgence ». Dès 2014, la préconisation d'un renforcement durable de la participation de l'État dans le financement de l'APA et la réévaluation tarifaire du service rendu par les associations d'aide à domicile étaient donc Les structures réunies la semaine dernière nous ont rappelé qu'il existe dix-sept diplômes ou intitulés de postes différents pour une même réalité. Les droits et avantages de tous ces salariés varient en fonction des conventions collectives, ce qui provoque une volatilité des compétences et des savoir-faire dommageable, en premier lieu, aux personnes accompagnées. Il y a urgence à constituer un véritable service public national de l'autonomie et du grand âge. Nous devons élever la qualité du service rendu à la personne âgée et permettre une réelle reconnaissance de la profession.

employeurs ne contribueront qu'à hauteur de 6 % au soutien à l'autonomie. Pour notre part, nous considérons que les dépenses liées à la perte d'autonomie doivent relever de la branche assurance maladie de la sécurité sociale. De même, soumettre les revenus financiers des entreprises à des cotisations sociales modulées selon la politique salariale et environnementale permettrait de recruter 100 000 personnels à l'hôpital et 100 000 personnels par an pendant trois ans au profit des Ehpad et du secteur médico-social. La taxation des laboratoires pharmaceutiques et des Ehpad privés lucratifs permettrait également d'assurer la création d'un pôle public du médicament, des dispositifs médicaux et de la recherche. Afin de regagner notre souveraineté sanitaire et de lutter contre les pénuries de médicaments, il est indispensable que nous regagnions en 2021 des capacités de production et de distribution des médicaments ou des vaccins. Nous aurions apprécié de trouver dans ce texte de vraies propositions pour lutter contre la désertification

pour favoriser l'installation de jeunes médecins et en former un plus grand nombre dans les facultés. Ce PLFSS est le dernier de votre gouvernement. Pourtant,

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 subit l'impact simultané de l'agenda politique et de la crise sanitaire et économique. Je remercie la rapporteure générale et les rapporteurs thématiques de la qualité de leurs rapports, qui éclairent avec précision et mise en perspective ce texte, je salue l'acuité du regard que mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe porte sur les enjeux financiers de ce PLFSS. Je souhaite aborder plus particulièrement la branche autonomie, qui ne vit pas ses meilleurs jours après la crise traversée par le secteur médico-social. Si l'on peut reprocher à ce PLFSS un manque de vision d'ensemble, les quelques dispositions qui s'y trouvent nous semblent de bon sens : mise en oeuvre des mesures du Ségur de la santé, amélioration de la prévention et de l'accès aux soins, lutte contre l'obésité infantile, actions de soutien à l'innovation pharmaceutique ainsi qu'à la perte d'autonomie, ou encore renforcement de la médicalisation des Ehpad et des liens avec les services d'aide à domicile. Néanmoins, les sénateurs du groupe Union Centriste regrettent profondément que la réforme ambitieuse pour le grand âge ne cesse d'être reportée depuis quinze ans. À l'annonce récente de la non-programmation d'une loi dédiée au cours de ce quinquennat, les professionnels des établissements, les services pour personnes âgées et les associations ont ressenti « un sentiment d'abandon

et ambitieux. Nous devons présenter des mesures fortes et concrètes pour réformer durablement l'accompagnement des personnes âgées ainsi que la qualité de vie au travail des professionnels du secteur. Il était ainsi attendu que le Gouvernement muscle le volet grand âge du PLFSS en intégrant les mesures les plus urgentes concernant la gouvernance et le financement de l'autonomie, des mesures essentielles pour un secteur qui se trouve dans une situation d'extrême difficulté. Les annonces de crédits supplémentaires en 2022 pour l'aide aux personnes âgées, notamment dans le secteur de l'aide à domicile, sont intéressantes, mais elles ne sauraient constituer une réponse suffisante à l'urgence de la situation, tout particulièrement dans le secteur des Ehpad. L'objectif de dépenses de la branche autonomie pour 2022 s'élève à 34,2 milliards d'euros. Cette somme finance essentiellement deux nouveautés : des revalorisations salariales issues du Ségur de la santé et un tarif plancher national pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). On ne peut que s'en féliciter.

Le Gouvernement propose également la généralisation des infirmières de nuit ainsi qu'une légère augmentation du temps de travail du médecin coordinateur en Ehpad. Néanmoins, ces annonces, souvent faites sans aucune concertation préalable, ni avec les professionnels ni avec les départements, ne sont pas en mesure de pallier l'absence criante d'une vision pluriannuelle. En ce qui concerne le handicap, je regrette que l'Assemblée nationale ait rejeté le principe de l'individualisation du calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), proposé par le sénateur Philippe Mouiller à travers une proposition de loi. Je déplore aussi que le groupe de travail qui devait être mis en place depuis deux ans sur l'accessibilité des transports pour les personnes en situation de handicap n'ait pas vu le jour. Cependant, j'apprécie que l'allocation journalière du proche aidant soit élargie et indemnisée au SMIC pour les « proches aidants de personnes dont le handicap ou la perte d'autonomie peuvent, sans être d'une particulière gravité, nécessiter une aide régulière ». La même revalorisation sera appliquée à l'allocation journalière de présence parentale. cette mesure est loin d'être satisfaisante. Moins de 5 000 personnes en ont bénéficié jusqu'à présent. Cette proposition reste au milieu du gué et ne répond pas à une demande exprimée de longue date date : son élargissement aux aidants dont les proches souffrent de longues maladies, notamment de cancers, afin que davantage de personnes puissent soutenir un proche malade nécessitant un accompagnement important. Les personnes malades relèvent de votre champ de compétence, monsieur le ministre. Pourquoi ne pas agir pour soutenir leurs proches aidants ? Par ailleurs, je propose que la différence entre l'allocation du proche aidant et le salaire puisse être couverte par les contrats collectifs de santé, en assortissant cette

Adoptée dans le cadre du pacte de refondation des urgences et dans le PLFSS pour 2020, cette mesure vise à élargir le cadre de cette pratique en ville afin de limiter le recours aux urgences pour des besoins d'examens de biologie de routine. Elle favorise, comme alternative aux passages aux urgences, l'accès des patients à ces examens. Force est de constater que ce service de proximité n'est toujours pas une réalité pour nos concitoyens. Il est incompréhensible que, deux ans après le vote de cette mesure, il n'existe toujours aucun travail publié au niveau réglementaire par le ministère. Il semble que la difficulté provienne de la négociation tarifaire de la CNAM pour coter l'acte de biologie délocalisé. Face à l'urgence de la situation, quand pourrez-vous enfin proposer ce modèle aux biologistes médicaux dans les établissements de santé, les maisons de santé ou les Ehpad ? L'article 42 du PLFSS pour 2022 propose la généralisation d'expérimentations dans le domaine de la santé. Je m'interroge sur la raison pour laquelle le Gouvernement n'a pas souhaité généraliser l'expérimentation du dépistage du virus de l'hépatite C, alors qu'il s'est fixé, dans le cadre du plan national Priorité prévention » de 2018, l'objectif ambitieux d'élimination de ce virus en France à l'horizon de 2025. Je me réjouis du remboursement des moyens de contraception accordé aux femmes jusqu'à l'âge de 25 ans. Il s'agit d'une avancée majeure pour toutes, mais pas pour tous Alors que la charge contraceptive concerne autant les femmes que les hommes, l'annonce du Gouvernement apparaît comme un rendez-vous manqué, puisqu'elle oublie la contraception masculine et, surtout, la place des hommes dans le partage de la contraception. Il est temps de les impliquer davantage En ce qui concerne les sages-femmes, il est nécessaire de répondre de manière pertinente à leurs revendications, lesquelles me semblent bien légitimes. C'est un sujet qui mérite votre attention, monsieur le ministre.

Cette disposition n'a pas sa place dans le code de la santé publique ; une telle inscription n'est ni rigoureuse ni sérieuse. Les préoccupations légitimes de ces personnels méritent une réponse d'apaisement, des actions concrètes, et non une disposition législative qui sera assurément retoquée par le Conseil constitutionnel. bien sûr important de faire connaître les compétences des sages-femmes, et une campagne d'information permettra d'améliorer l'accès aux soins des femmes sur nos territoires. Vous savez que le Sénat est sensible à ce sujet. En revanche, l'article 34 de la Constitution ne prévoit pas que la loi soit le support marketing de la communication gouvernementale Aussi, nous voterons l'amendement de suppression proposé par Mme la rapporteure. Permettez-moi de conclure par un proverbe anglais : « un homme qui promet beaucoup et qui ne tient rien ressemble à un jardin où il ne pousse que de mauvaises herbes. » Il suffit de ne pas multiplier les promesses, si vous n'êtes pas en mesure de les concrétiser. Notre message est clair : vos efforts ne sont malheureusement pas à la hauteur des attentes, malgré la création d'innombrables missions et groupes de travail dont peu d'enseignements sont tirés pour faire progresser la prise en charge des plus fragiles. La parole est à Mme

dont la vie ne peut se dérouler sans l'aide de proches ou de professionnels, ainsi que la carrière de celles et ceux qui les accompagnent, et dont c'est le métier.

puis aux liens entre les générations, n'a finalement rien proposé du tout. Ces effets d'annonce n'ont eu pour conséquence que d'amplifier le désarroi

décriée par tout le secteur. Elle est considérée comme étant pénalisante pour les départements bons élèves. Vous y avez ajouté un bonus qualité complémentaire allant jusqu'à 3 euros, soit un reste à charge plus important, donc plus lourd pour les plus modestes. Ainsi, vous creusez un peu plus encore les inégalités. La France est en retard dans la prise en charge de la dépendance et du handicap ; en retard sur la prévention de la perte d'autonomie. Pourtant,

premièrement, la préservation des droits à la retraite des indépendants travaillant dans les secteurs les plus touchés par la crise. Ainsi, certains d'entre eux n'ont pu valider leurs trimestres de retraite durant la crise sanitaire en raison du ralentissement, voire de l'arrêt de leur activité. effet collatéral est corrigé par le projet de loi : désormais, les indépendants les plus touchés par la crise bénéficieront d'un nombre de trimestres de retraite validés en 2020 et 2021 équivalent à la moyenne des trimestres validés lors de leurs trois derniers exercices.

Je pense notamment au recrutement de personnels dans les centres médico-psychologiques (CMP) pour les adultes et les enfants, mais aussi au déploiement d'un service téléphonique d'accès aux soins psychiatriques

S'agissant des pénuries de médicaments, dont nous aurons, je l'espère, largement l'occasion de parler ces prochains jours, un amendement des députés durcit les sanctions contre les mauvaises pratiques de certains grossistes répartiteurs, dits, qui ne respectent pas leurs obligations de service public, en particulier celles de disposer d'un stock de médicaments et d'être en mesure de livrer les pharmacies dans un délai de vingt-quatre heures. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont permis l'expérimentation, dans six départements, d'un accès direct, sans ordonnance, aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes exerçant dans des structures de soins coordonnés.

Cette mesure concrète offre un meilleur accès aux soins et une véritable réduction des délais d'attente. En revanche, pour se prémunir d'une dégradation de la prise en charge des patients, la commission des affaires sociales souhaite garantir des « critères exigeants » dans la réalisation des bilans par les orthoptistes. Les textes d'application devront être pris après l'avis du Conseil national professionnel d'ophtalmologie. La commission exige également que les bilans visuels ne concernent qu'une tranche d'âge particulière, afin notamment de « prévenir les pertes de chance pour les patients les plus âgés Fruits du bicamérisme, ces mesures concrètes amélioreront le quotidien de milliers de personnes. Dans ce contexte de pandémie qui nous oblige, plusieurs autres défis doivent être relevés par ce PLFSS. Je ne doute pas que nos débats apporteront certaines améliorations. Je compte sur vous non seulement pour ne pas faire l'impasse sur la maîtrise de nos dépenses, mais également pour renforcer nos outils de régulation. La parole est à Mme Florence

est le dernier du quinquennat ; il est aussi celui de la sortie de la crise sanitaire. Malgré un budget de plus de 500 milliards d'euros, ce texte reste très en deçà des attentes des Français et des professionnels du secteur médical. Je ne reviendrai pas sur les observations de notre collègue Chantal Deseyne, auxquelles je souscris pleinement ! Monsieur le ministre, face à la pandémie de covid-19, notre système de santé n'a tenu que grâce au dévouement et à la compétence des personnels soignants. Certes, il y a eu le Ségur de la santé, mais tous les professionnels ne sont pas concernés par les augmentations de salaire prévues. Il y Il y a les nombreux oubliés, qui, pourtant, n'ont pas ménagé leur peine depuis le début de la crise sanitaire ! Et il y a aussi tous les déçus de vos propositions, qui consistent en des effets d'annonce. Les sages-femmes, les infirmiers, les médecins, les pédiatres, les ophtalmologistes, les psychologues : la liste des insatisfaits est longue. Le Gouvernement fait montre de bien peu de considération et de reconnaissance envers ces professions. Ben voyons ! En premier lieu, je pense aux sages-femmes, grands oubliés du Ségur. La France compte environ 23 000 sages-femmes en activité, dont 97 % sont des femmes. Celles exerçant à l'hôpital bénéficieront à partir de janvier d'une prime de 100 euros et d'une hausse de salaire d'environ 100 euros brut par mois. Malgré cela, les niveaux de rémunération restent inadaptés à leur niveau de responsabilités.

et non plus seulement d'un médecin. Il prévoit également des campagnes de communication organisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour informer la population sur leurs compétences ! C'est stupéfiant ! J'en viens à un autre sujet de mécontentement : de la construction d'une psychiatrie humaine ? L'état psychiatrique du pays s'est aggravé avec la crise sanitaire et, là encore, les besoins sont criants. Alors que les maladies psychiques touchent chaque année une personne sur cinq, soit 12 millions de Français, dont seuls 40 % à 60 % d'entre eux sont pris en charge, ce PLFSS ne comporte aucune mesure nouvelle pour la psychiatrie et la pédopsychiatrie. Actuellement, 30 % des postes de praticiens hospitaliers sont vacants dans le public, compte tenu du niveau des salaires et de la détérioration des conditions de travail. En outre, la psychiatrie ne séduit plus les étudiants, puisque ceux-ci boudent plus de 10 % des postes d'internat de cette spécialité. Présenté comme la mesure phare des assises de la santé mentale, le remboursement des consultations de psychologues ne rencontre pas le succès escompté auprès des professionnels du secteur. Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de cette mesure sont en décalage complet avec la pratique des consultations des psychologues. Nous essaierons néanmoins d'améliorer ce dispositif en séance. Notre collègue Alain Milon développera tout à l'heure la situation de la psychiatrie en France dans son intervention. La pédiatrie est un autre secteur en grande difficulté. Huit départements connaissent une densité inférieure à un pédiatre pour 100 000 habitants et l'âge moyen des pédiatres libéraux laisse présager une aggravation de la situation, puisque 44 % d'entre eux ont plus de 60 ans. Cette situation pose une question majeure d'accès aux soins pédiatriques. Mais ce PLFSS ne formule aucune proposition. Monsieur le ministre, nous attendions des mesures fortes en direction des soignants pour corriger tous les manquements du passé. Au lieu de cela, le Gouvernement nous offre des rustines ! Pis encore, une nouvelle étape est franchie dans le démantèlement des compétences médicales, avec un risque important de dégradation de la qualité des soins.

Abandonner les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les sages-femmes revient à abandonner ceux qui luttent au quotidien pour préserver la santé de tous nos concitoyens ! Nous plaidons pour une réelle politique d'attractivité des métiers de la santé et du social, avec des rémunérations de base attractives qu'une meilleure évolution des carrières et des salaires. Malheureusement, le droit d'amendement ne nous permet pas de faire des propositions en ce sens. Nous comptons néanmoins sur des échanges constructifs avec le Gouvernement pour améliorer ce PLFSS, et nous espérons, messieurs les ministres, que vous accepterez de lever certains gages sur nos propositions d'amendements

Avant même la crise sanitaire, en janvier 2020, plus de 1 500 médecins démissionnaient de leurs fonctions d'administration, de gestion et de représentation pour protester contre le refus du Gouvernement de négocier avec les parties prenantes sur les moyens de l'hôpital public. Le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale de la mandature n'est pas à la hauteur dans ces deux domaines, ni dans d'autres au demeurant. C'est en effet un « presque » qu'inspirent les diverses mesures mises en avant dans ce texte : de nombreuses dispositions, à première vue prometteuses, ne vont pas jusqu'au bout de ce qui peut être proposé. Si l'on peut ainsi saluer certaines mesures intéressantes, telles que la gratuité de la contraception jusqu'à 25 ans, ou la généralisation de l'intermédiation pour le versement des pensions alimentaires,

la fluidité de la transmission des informations entre administrations et organismes n'est pas garantie. Enfin, ces prestations sont des droits quérables, qui nécessitent de la part des bénéficiaires potentiels de mener à bien un certain nombre de démarches identifiées comme favorisant le non-recours.

cumulant les supposés inconvénients du salariat, notamment le lien de dépendance vis-à-vis de l'entreprise, avec ceux du véritable travail d'indépendant, notamment en ce qui concerne l'accès à la protection sociale. Nous refusons d'emprunter ce chemin, et demeurons attachés à la préservation d'un authentique salariat et d'un véritable statut d'indépendant. Nous y reviendrons très vite avec l'examen du projet de loi de ratification de l'ordonnance relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes.

Nous avons pris bonne note que le Gouvernement a peu à peu rectifié le tir. Je pense notamment à l'amendement au PLFSS 2021 qui a concrétisé un avenant à leur convention collective de branche. Mais les modalités de répartition de cette revalorisation appliquée au 1 octobre n'ont pas fait l'unanimité, une partie des salariés du secteur en étant de fait exclue.

Dans ces conditions, l'article 30 du PLFSS, qui prévoit de consolider le financement des SAAD avec un tarif plancher national de 22 euros par heure, est certes intéressant, mais il ne peut pallier une politique structurellement insuffisante en la matière,

entrée en vigueur le 1 octobre dernier, s'élèverait à 75 millions d'euros en 2021, compensé par l'État à hauteur de 70 %, par l'intermédiaire de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le coût résiduel pour les départements serait de 22 millions d'euros, l'État s'engageant à couvrir 50 % de la dépense supplémentaire à partir de 2022, pour un montant total de 150 millions d'euros. de rappeler que, désormais, les départements ne disposent plus de l'autonomie fiscale. Il faudrait s'en souvenir au moment de décider le déploiement de mesures les mettant à contribution, alors même qu'ils n'ont plus les moyens d'ajuster les recettes aux nouvelles dépenses qui leur sont imposées dans votre propos liminaire que le Gouvernement confirmait le virage « domiciliaire ». Mais où sont les financements ? Il serait illusoire de penser que les mesures dont je viens de parler seront suffisantes. des retraites, si le Gouvernement propose des mesures fonctionnelles, dont certaines vont dans le bon sens, comme la retraite progressive étendue aux cadres, nous ne sommes pas dupes Bien que vous n'ayez finalement pas mené à bien la réforme envisagée, nous sommes sur la défensive, tant les atermoiements ont été nombreux à ce sujet. Je sais bien que le Gouvernement- et il n'est pas le seul -attend le moment opportun pour imposer des réformes qui seront contraires aux intérêts du plus grand nombre de salariés. J'entends ici et là que les seules solutions consisteraient à ajouter des trimestres et à reporter l'âge de départ, et donc à faire toujours payer les mêmes catégories de travailleurs : nous nous y opposerons. Les avancées sociales mises en avant par ce PLFSS dissimulent le refus de mener les politiques publiques nécessaires à la préservation et à la modernisation de notre modèle social. Le quinquennat qui se termine - entre la crise des « gilets jaunes » et les fragilités que la covid-19 a mises en avant Nous aurions pu espérer un PLFSS de combat, mais il s'agit d'un texte de routine. Cela me semble d'autant plus surprenant que, depuis quelques jours, les ministres se succèdent dans les médias pour se réjouir d'une situation économique qui connaîtrait une embellie. Se pose donc la question de la répartition des bénéfices de cette sortie de crise. Iront-ils à l'hôpital public, à l'autonomie ? Ce ne sera- hélas ! -pas le cas

l'examen du PLFSS 2022 m'offre l'occasion de vous alerter sur la situation très préoccupante de la psychiatrie publique en France. En 2019, les professeurs Marion Leboyer et Pierre-Michel Llorca ont coécrit

aux difficultés structurelles de la fonction publique hospitalière. En outre, l'application discriminante de certaines mesures a généré incompréhension, frustration et colère chez certains professionnels.

Cette sous-évaluation porte sur le complément de traitement indiciaire et sur la revalorisation de traitement des personnels médicaux. il existerait un différentiel de 15 % à 20 % des crédits alloués par établissement. Cet écart s'explique essentiellement par le fait que ces mesures ont été calculées sur le fondement de

À cela s'ajoute la pénurie médicale, qui touche tous les établissements publics de santé, mais surtout certaines spécialités, dont les plus concernées sont les urgences, la réanimation, la gynécologie et la psychiatrie. Les établissements de santé plaident de longue date pour un contrôle et une régulation ferme du marché de l'intérim médical, et nous adhérons à la philosophie de la loi du

qui subit des démissions d'intérimaires médicaux, la mise à mal de la permanence des soins et des fermetures de lits ou de services. Les sommes exorbitantes consacrées à l'intérim médical

alors qu'un intérimaire en psychiatrie gagne entre 600 et 850 euros net par jour, soit 13 000 euros net par mois. La rémunération des intérimaires médicaux est immorale et indécente. Des établissements de santé mentale de ma région sont fortement touchés par cette situation, au risque de devoir revoir à la baisse les capacités d'hospitalisation complète, alors que la demande de la patientèle augmente.

soit de patients suivis de longue date, pouvant faire des épisodes délirants aigus qui nécessitent des traitements de crise. Cette population peut être à la fois malade et délinquante, avec des degrés de dangerosité variable. Ces situations complexes supposent des parcours de soins fluides et réactifs entre établissements de santé ayant des structures spécialisées, mais également une articulation entre la justice, la police et l'hôpital. Les députés ont de nouveau voté le renforcement du contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD) sur les pratiques d'isolement et de contention en psychiatrie, prévu à l'article 28 du PLFSS 2022. En juin 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que les mesures d'isolement et de contention en milieu psychiatrique constituent une privation de liberté, et les a déclarées contraires à la Constitution, au motif que le législateur n'avait pas fixé de limite à la durée de ces mesures. Les effets de cette abrogation ont été reportés au 31 décembre 2020. Le Gouvernement a alors pris des mesures correctrices dans le PLFSS pour 2021. Celles-ci ont été de nouveau partiellement censurées, avec un effet différé au 31 décembre 2021.

L'instauration de cette mesure aurait considérablement alourdi le travail des JLD et « technocratisé » les procédures au sein des établissements. En effet, ce contrôle s'appliquerait dès la seconde période de douze heures d'isolement ou de six heures de contention.

pour créer des zones d'apaisement dans les services. Le respect des droits fondamentaux des patients placés sous le contrôle du JLD ne doit pas engendrer un accroissement de l'insécurité pour la société. Certains patients ont besoin, cliniquement, de temps d'isolement.

pour malades difficiles (UMD) ou d'une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) pour recevoir des personnes incarcérées nécessitant des soins psychiatriques. L'UHSA de Marseille n'est que partiellement ouverte depuis 2018 ; il y manque encore 20 places. L'accès L'accès aux UMD est de plus en plus difficile sur l'ensemble du territoire national. L'articulation clinique avec les services demandeurs est lacunaire et les sorties unilatérales mettent en difficulté les équipes médicales et paramédicales, lorsque celles-ci doivent recevoir dans l'urgence des patients dangereux. L'irresponsabilité pénale est un sujet délicat qui resurgit à l'occasion de faits divers dramatiques, mais il faut être conscient que l'auteur de faits criminels peut passer un an et demi en détention provisoire. Après avoir été déclaré irresponsable pénalement, ce même individu peut passer d'un centre pénitentiaire à un centre hospitalier spécialisé ouvert, sans que les soignants qui l'accueillent connaissent ni son dossier pénal ni sa dangerosité.